La séance est reprise.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai l'honneur de vous présenter le projet de loi de finances pour 2021 tel qu'il a été adopté, il y a quelques jours, par l'Assemblée nationale.

L'accord trouvé en commission mixte paritaire permet d'envisager l'adoption et la mise en oeuvre de ce texte dans les meilleurs délais. Ainsi, face à cette crise épidémique et économique sans précédent, le Gouvernement a mis en oeuvre une réponse massive.

Nous avons mis en place un dispositif de financement de l'activité partielle à un niveau inédit pour ce qui nous concerne et inégalé sur la scène européenne. Ce faisant, nous avons pu prendre en charge jusqu'à 12 millions de personnes lors du premier confinement. Nous avons mis en place un fonds de solidarité, aujourd'hui bien connu, qui a profité à plus de 2 millions d'entreprises et dont les critères ont été revus à l'aune des débats parlementaires et de diverses contributions.

Dans ce contexte, le projet de loi de finances pour 2021 revêt une importante particulière. Il doit permettre au Gouvernement de donner à notre pays les moyens de la relance économique, pour le sortir de la crise, de tenir ses engagements et de financer ses priorités. Il doit également prendre en compte, en suivant un double objectif de sincérité budgétaire et de réalisme économique, les dernières évolutions de la pandémie et ses conséquences sur nos hypothèses macroéconomiques comme sur la trajectoire des finances publiques.

». De plus, parmi ces 16,5 milliards d'euros, un certain nombre de crédits ont déjà fait l'objet d'une adoption par le Parlement. Je pense aux dispositifs de soutien aux collectivités territoriales et notamment

une dizaine de milliards d'euros au titre de 2020 et une quarantaine de milliards d'euros au titre de 2021, par le truchement des missions et des opérateurs que j'ai évoqués.

Enfin, ce projet de loi de finances comporte un certain nombre de mesures relevant de réformes structurelles comme la mise en oeuvre- enfin ! diront certains -de la contemporanéisation de (APL). Je pense également à la facturation électronique que nous proposons de rendre obligatoire à compter de 2023, afin d'améliorer nos possibilités de lutte contre la fraude fiscale, notamment en matière de carrousels de TVA.

nous vous l'avons indiqué lors des débats sur le PLFR 4 et à l'occasion de l'actualisation des sous-jacents du PLFSS, nous avons corrigé nos hypothèses macroéconomiques pour 2020.

-et le poids de la dette publique de 117,5 % à 119,8 % du PIB. Ces chiffres sont, aux yeux d'autres analystes, particulièrement prudents, la Banque de France et l'Insee considérant dans leurs propres travaux

le choix de la prudence pour nos hypothèses. Le Haut Conseil des finances publiques a toujours qualifié les hypothèses de travail du Gouvernement de « plausibles et prudentes » ou de « plausibles, mais prudentes ». Nous avons donc à réviser un certain nombre de sous-jacents des textes que nous vous présentons.

le texte a évidemment évolué lors de son examen par l'Assemblée nationale et, si le temps ne me permet pas de revenir en détail sur chacune des dispositions initialement prévues, je tiens à souligner que l'Assemblée nationale l'a enrichi de nombreux amendements, près de 400 ayant été adoptés.

la rénovation du dispositif de péréquation régionale conformément à l'accord signé par le Premier ministre avec les présidents de région le 28 septembre dernier ; la modification des critères d'attribution du fonds de stabilisation pour les départements, pour qu'il puisse bénéficier à une cinquantaine de départements au lieu de trente auparavant, et alors qu'il est porté à 200 millions d'euros au lieu de 115 millions habituellement. L'Assemblée nationale a, enfin, adopté les amendements visant à faciliter la mise en oeuvre du plan de relance, notamment en permettant des dépenses anticipées sur un certain nombre de sujets.

pour les rendre plus justes et plus efficients. Enfin, en cohérence avec la proposition du Gouvernement que j'ai évoquée, ils ont créé un dispositif de soutien aux entreprises locataires de moins de 5 000 salariés pour leur permettre de faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Il permet la prise en charge par l'État d'une partie des loyers, sous la forme d'un crédit d'impôt accordé aux bailleurs égal à 50 % des loyers abandonnés normalement dus au cours de la période d'application des mesures de confinement pour les entreprises de moins de 250 salariés, et à 33 % pour les entreprises d'une taille supérieure. L'ensemble des amendements adoptés par l'Assemblée nationale conduit évidemment à une dégradation du solde budgétaire de 344 millions d'euros par rapport au point d'entrée en discussion. Ce solde budgétaire s'établirait à 153,1 milliards d'euros en 2021, déficit exceptionnellement élevé qui traduit l'impact de la crise sur les finances publiques et la mise en oeuvre du plan de relance. Pour conclure, nous proposons, comme je vous l'ai dit, une révision des hypothèses macroéconomiques au fil de l'eau, avec un objectif de sincérisation des textes et d'adoption de la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances pour 2020 avec les mêmes hypothèses, les mêmes sous-jacents et la même trajectoire macroéconomique. Nous sommes en mesure de le faire pour 2020 et nous vous proposons de faire de la même manière pour 2021.

relativement fort, facteurs qui ont d'ailleurs expliqué la forte reprise du troisième trimestre. Toutefois, la recrudescence de l'épidémie cet automne montre que sa maîtrise sera plus exigeante cet hiver. Aussi avons-nous intégré à nos projections de croissance des comportements plus prudents de la part de tous les acteurs. Nous avons ainsi proposé au Haut Conseil des finances publiques de chiffrer le rebond de l'activité l'année prochaine à 6 % au lieu de 8 %, toujours mobilisés par la mise en oeuvre du plan de relance que nous sommes en train de déployer. La révision du scénario macroéconomique et cette hypothèse de croissance à 6

pour tirer les conséquences de cette révision dans le PLF et modifier l'article liminaire pour la prévision relative à 2021. Mais nous le ferons, si vous en êtes d'accord, dans un instant, pour la prévision

les bonnes solutions en matière de gouvernance, de définition de trajectoire pluriannuelle des finances publiques, de maîtrise et de cantonnement de la dette, d'amélioration des processus d'élaboration de la décision budgétaire et, peut-être, de perspectives pluriannuelles en la matière.

de la discussion générale sur le projet de loi de finances pour 2021. J'ai la conviction que les échanges qui vont nous réunir pendant plusieurs jours constitueront autant d'occasions de continuer à améliorer ce texte et, je l'espère, à trouver de grandes convergences. La parole est

alors, de retrouver des marges de manoeuvre budgétaires, tant que les indicateurs économiques étaient au vert, pour se préparer à l'éventualité d'une nouvelle crise. Eh bien, malheureusement, nous y sommes ! L'épidémie de covid-19 a tout bouleversé sur son passage : trois lois de finances rectificatives, bientôt quatre, ont été votées, y compris, en pour que les entreprises, les ménages et les collectivités territoriales soient soutenus pour traverser cette terrible période. Il y a quelques semaines encore, le PLF pour 2021 devait être celui de la relance, mais avec le rebond de l'épidémie et la décision de reconfinement national, les priorités ont de nouveau changé. Nous venons ainsi d'apprendre que le Gouvernement prévoit de réviser le taux de croissance pour 2021 de 8 % et que les dispositifs d'urgence devraient évoluer d'ici quelques semaines, pour être intégrés dans le projet de loi de finances. Autrement dit, nous discutons d'un texte qui pourrait, sous peu, ne plus ressembler à ce qu'il est aujourd'hui. Par respect

En pareilles circonstances, ce manque de respect est une faute ! Revenons-en au texte qui nous est transmis. L'économie française a bien résisté au choc du premier confinement, grâce, notamment, aux mesures de soutien que nous avons adoptées et qui ont pu à la fois préserver les revenus des ménages et, dans une moindre mesure, des entreprises. Le rebond en sortie de confinement a été rapide, avec une hausse du PIB de 18,2 %. Dans ce contexte, le Gouvernement a annoncé, au début du mois de septembre, un plan de relance indispensable pour aider l'économie à surmonter la crise. Ce plan de relance me paraît bien calibré en termes de montant, même s'il faut relativiser les 100 milliards d'euros puisque, en particulier, sont pris en compte 15 milliards d'euros de mesures déjà engagées en 2020, que le montant de la baisse des impôts de production y est compté deux fois et sans tenir compte de l'« effet retour » de l'impôt sur les sociétés. Si le montant global est donc satisfaisant, les mesures et le calendrier retenus ne répondent en revanche que très imparfaitement aux critères d'efficacité d'un « bon » plan de relance. En effet, pour être efficace, un plan de relance doit être mis en oeuvre rapidement, composé de mesures temporaires et avoir un fort effet multiplicateur sur l'activité à court terme. Aucun de ces trois critères n'est véritablement rempli. Le plan de relance est avant tout trop tardif, comme l'illustre la comparaison avec l'Allemagne. Si le montant des deux plans est comparable, la quasi-totalité du plan de relance allemand devrait avoir été déployée d'ici à la fin de l'exercice 2021, contre, à la même époque, seulement la moitié du plan français. Ce plan de relance aura par ailleurs un effet modéré sur la croissance en 2021, estimé entre 1,1 et 1,2 selon les estimations. De même, un cinquième du plan de relance correspond à des mesures permanentes qui pèseront durablement sur les comptes publics, ce qui, là encore, est problématique. Je souligne et regrette les grandes insuffisances du plan de relance initial à l'égard des plus fragiles qui sont les grands oubliés, notamment en comparaison avec le plan Sarkozy adopté lors de la crise de 2009. Si le plan de relance initial me semblait donc déjà mal calibré, le reconfinement va naturellement imposer de renforcer la logique de soutien. De ce point de vue, nous souhaitons que le plan de relance comprenne davantage de mesures de renforcement des fonds propres des entreprises et de soutien aux personnes précaires, comme aux collectivités territoriales. Une nouvelle fois, votre plan est trop administré depuis Paris, malgré vos tentatives de déconcentration. Monsieur le ministre, appuyez-vous sur les élus locaux qui savent, mieux que d'autres, mobiliser les énergies pour relancer l'activité sur leurs territoires. En tout état de cause, votre scénario budgétaire pour 2021 apparaît sérieusement compromis par le reconfinement. Dans un scénario intermédiaire fondé sur une croissance de 6 % et 15 milliards d'euros de soutien supplémentaire, nous estimons que le déficit atteindrait 8,6 % du PIB et la dette 122,3 % du PIB à l'issue de l'exercice 2021.

Mais au-delà de l'évolution de court terme de la trajectoire budgétaire, il ne faut pas perdre de vue l'impact qu'auront ces décisions sur l'état de nos finances publiques à moyen terme. Or, de ce point de vue, la cote d'alerte est atteinte et il faut impérativement privilégier les mesures temporaires, puissantes et bien ciblées, pour favoriser la sortie de crise. En effet, celle-ci s'accompagne, avec votre budget, de hausses de dépenses et de baisses de recettes pérennes que nous estimons à 45 milliards d'euros sur la période 2020-2024. Au total, le déficit structurel français devrait dépasser 5 % du PIB en sortie de crise. Concrètement, il faudra déjà réaliser environ 75 milliards d'euros d'économies en sortie de crise, uniquement pour ramener le déficit structurel à son niveau de 2019, ce qui est encore ce qui est encore trop élevé pour réduire significativement l'endettement que notre pays porte comme un fardeau trop encombrant. Une fois la crise surmontée, la France devra retrouver des marges de manoeuvre budgétaires, afin d'éviter que la faiblesse de la croissance, conjuguée à une hausse du coût de financement, ne fasse basculer l'économie dans une spirale négative, comme en Italie. Ramener l'endettement autour de 100 % du PIB d'ici à 2030 pourrait ainsi constituer un objectif central, dès lors que l'on compte une crise tous les cinq à dix ans en moyenne. S'agissant du budget de l'État proprement dit, le déficit est pour le moment prévu à 153 milliards d'euros dans le projet de loi de finances, en baisse par rapport à 2020. Quels en sont les déterminants ? Tout d'abord, les dépenses du plan de relance en 2021 seraient moins élevées que celles du plan d'urgence en 2020. Ensuite, les recettes rebondiraient après leur chute de cette année et le budget bénéficierait des premiers versements du plan de relance européen. Mais tout ceci est encore bien incertain Certes, la charge de la dette reste à un niveau historiquement bas, mais ne nous y trompons pas : l'État doit à la fois payer les dépenses budgétaires de l'année et renouveler une dette considérable qui vient de dépasser le seuil des 2 000 milliards 2 000 milliards d'euros par l'accumulation de quarante-cinq années de déficits. Soulignons que l'État se finance désormais autant par l'endettement que par l'impôt. Si les taux remontaient, l'impact serait considérable et durable, et l'effort pourrait devenir insurmontable. Je ne commenterai pas le niveau attendu des recettes, car il est, à l'heure actuelle, trop incertain, les hypothèses du projet de loi de finances étant déjà dépassées. Je rappellerai simplement les transformations importantes qu'elles connaissent une nouvelle fois cette année, compte tenu des réformes des impositions locales qui entraînent l'affectation de nouvelles parts de TVA aux collectivités. Les dépenses de l'État progressent fortement sans qu'elles soient toutes nécessairement liées à la crise. De votre vaste programme de réformes de structure intitulé Action publique 2022, il ne reste presque plus rien, en particulier en matière de réduction de l'emploi public. Mais soyons clairs, les crises, qu'elles soient sanitaires, sociales, comme celle des « gilets jaunes », ou environnementales, risquent de se renouveler avec un possible effet amplificateur. Loin d'attendre un retour hypothétique à la normale, il faut que l'économie soit capable de s'adapter à ce monde nouveau. À ce titre, la réponse à la crise environnementale devient urgente et nécessitera une prise en compte et des décisions fortes et courageuses s'inscrivant dans le long terme. La relance de l'économie doit être mise à profit pour insuffler un renouveau, un changement profond des paradigmes de nos modèles de production et de développement, s'appuyant, pour en faire autant de chances et d'atouts, sur certaines contraintes écologiques et environnementales. Pour être acceptées, les politiques environnementales doivent intégrer et traiter les situations de précarité sociale, économique et territoriale.

à la fiscalité sur les produits énergétiques. Nous devons donc aider les ménages à adapter leur comportement ! Au-delà du plan de relance et de la réforme des impôts de production, le projet de loi de finances compte finalement assez peu de mesures d'ampleur. Quels changements souhaitons-nous apporter à ce texte ? En ce qui concerne la réforme des impôts de production, qui constitue la principale mesure de ce PLF, je souhaite, d'ores et déjà, indiquer que, si la commission des finances n'a pas globalement remis en cause les réductions d'impôts locaux proposées, c'est parce que les entreprises, en particulier dans le secteur industriel, doivent voir leur niveau d'imposition se réduire pour rester compétitives. Mais il importe aussi d'assurer une juste et pérenne compensation aux collectivités territoriales. À ce titre, la commission des finances proposera que l'État compense, comme pour les régions, la perte de recettes de la cotisation sur la valeur

Vous y voyez un effet d'aubaine, nous y voyons un État qui revient sur sa parole, alors que cette mesure permet de couvrir les pertes de recettes et les hausses des dépenses des collectivités. La commission souhaite également, au nom de la solidarité nationale, que les assureurs versent une contribution exceptionnelle adossée à l'assurance dommages, compte tenu du faible taux de sinistralité enregistré pendant le confinement. ! Nous réfléchissons aussi à mettre en place une taxation exceptionnelle des grandes plateformes de la vente à distance, compte tenu de l'incroyable aubaine qui s'est offerte à elles avec la fermeture des commerces physiques et le confinement. Nos amendements complèteront également votre plan de relance pour qu'il puisse davantage porter ses fruits à court terme. Nous proposerons, notamment pour les entreprises, le report en arrière des déficits dans la limite de 5 millions d'euros, l'amélioration des coefficients d'amortissement dégressif, ainsi que des dispositifs spécifiques de suramortissement. Il faut aider les entreprises qui le peuvent à réaliser rapidement leurs investissements.

de soutenir nos compatriotes qui sont plus particulièrement touchés par la crise. Je pense tout d'abord aux travailleurs indépendants, à ces petites entreprises

Il faut également penser aux étudiants qui entrent sur le marché du travail, aux jeunes comme aux travailleurs plus âgés qui peinent à trouver un emploi. Les entreprises voudraient recruter, mais le contexte est difficile. Pour cela, nous proposons de prolonger le dispositif de prime à l'embauche pour six mois, en prévoyant qu'il s'applique aux PME pour les postes rémunérés jusqu'à 1,6 SMIC ou l'emploi de jeunes sans condition relative au salaire et avec une bonification. Enfin, il faut inciter les ménages et les entreprises à faire le pas de la transition écologique, sans tomber, bien sûr, dans la fiscalité punitive. C'est pour cela que je vous proposerai d'étaler sur cinq ans la hausse du malus automobile, tout tout en renforçant la prime à la conversion. Les entreprises doivent être soutenues dans cette démarche ; c'est pour cela que la commission des finances propose de faire passer d'un an à deux ans la durée du nouveau crédit d'impôt pour les travaux énergétiques dans les bâtiments tertiaires des PME. En conclusion, mes chers collègues, la commission des finances vous demande d'adopter les amendements qu'elle vous propose en attendant de savoir quelles seront les évolutions apportées à ce texte par le Gouvernement au cours des prochaines semaines. La parole

Le verbe « débuter » n'est d'ailleurs pas exact, puisque le marathon budgétaire a démarré dès le mois de septembre avec l'audition des ministres. Le rapporteur général, les rapporteurs spéciaux et les rapporteurs pour avis se sont mobilisés depuis plusieurs semaines pour étudier en détail ce budget.

J'en viens tout de suite aux principales caractéristiques de ce projet de loi de finances : un budget dit « de relance », mais qui est avant tout marqué par des incertitudes, des hésitations et quelques choix contestables. Je voudrais commencer par les incertitudes le cadrage macroéconomique qui nous est présenté est pour le moins mouvant et suit l'évolution de la situation sanitaire. Cette année a déjà été rythmée par quatre collectifs budgétaires et la situation est loin de se stabiliser. Le projet de loi de finances a été présenté au mois de septembre, au moment où il était question d'une offensive pour relancer l'économie, après une période estivale plutôt encourageante. Avec la décision d'un second confinement, un sérieux coup de frein a été donné. Désormais, le Gouvernement révise l'estimation de croissance à 6 % au lieu de 8 % pour 2021, tout en espérant, comme nous tous, pouvoir éviter un troisième confinement l'an prochain. Nous sommes, maintenant, bien loin du rebond présenté qui aurait pu, selon vous, nous permettre de retrouver dès 2022 notre niveau de richesse d'avant la crise. En termes d'hésitations, le ministre de l'économie annonce des mesures de soutien complémentaires à certains secteurs pour l'année 2021, mesures qu'il est en train d'examiner avec le Premier ministre et le Président de la République et qui, selon lui, seront décidées en fonction du calendrier sanitaire. Autant dire que nous débattons d'un texte provisoire, appelé, très rapidement, à de nouvelles corrections. Le Gouvernement donnera les chiffres révisés de déficit et de dette au début sans doute- mais cela nous a été confirmé -pour la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, alors que nous terminerons l'examen du PLF le 8 décembre. Dans le même temps, nous venons d'ouvrir des crédits en PLFR nous savons, d'ores et déjà, qu'une part considérable sera reportée, puisque pas moins de 47 programmes budgétaires, contre 20 l'an dernier, pourront faire l'objet de reports supérieurs à 3 % des crédits ouverts, ce qui brouille la lisibilité des exercices budgétaires. Quant à parler de la portée de l'autorisation parlementaire, je préfère passer d'aborder quelques choix contestables. Il ne s'agit pas de remettre en cause des mesures de soutien aux entreprises et à l'emploi,

La mission « Plan de relance », dotée, en 2021, de 36 milliards d'euros en autorisations d'engagement et de 22 milliards d'euros en crédits de paiement, prévoit également des moyens nouveaux, en particulier pour la rénovation énergétique, les infrastructures ou les énergies vertes. Mais elle recycle aussi beaucoup de mesures plus classiques qui auraient dû figurer dans les missions budgétaires : équipement des forces de sécurité, rénovation du patrimoine, transformation numérique des administrations publiques, etc. Par bien des aspects, ce plan est avant tout un plan de rattrapage. Il faudra juger de celui-ci sur ses effets concrets, car ce n'est pas tout d'ouvrir des crédits, il faut les consommer, si possible sur des projets porteurs d'avenir. Les crédits du plan de soutien sont loin d'être tous consommés cette année, qu'il s'agisse du fonds de solidarité ou des participations financières.

Le Gouvernement souhaite que le plan de relance soit temporaire, afin de ne pas grever durablement les finances publiques. Soit, mais comment expliquer alors que la baisse des impôts de production soit, elle, présentée comme pérenne ? le volet « cohésion » du plan de relance ne bénéficie pas de ce statut. Les plus démunis devront se contenter de mesures d'aide exceptionnelles et, pour tout dire, ponctuelles, qui ne sont malheureusement pas à la hauteur de la situation sociale de notre pays. Au sein du plan de relance, le volet « soutien aux personnes précaires » représente 86 millions d'euros. Nous savons tous aussi que le risque de paupérisation des jeunes exclus du marché du travail est bien réel. Si de nombreux leviers visant à la formation des jeunes ou à leur accompagnement vers l'emploi sont bienvenus, la période commande d'expérimenter sans délai une dotation pour l'autonomie de la jeunesse, qui permettrait à tous les jeunes émancipés de 18 ans à 25 ans de bénéficier de ressources pour se lancer dans la vie active. Ne tardons plus. Travaillons-y sans délai Il serait d'ailleurs invraisemblable que ce plan n'aide pas fortement ceux qui, demain, devront contribuer à le payer. Le PLF pour 2021 cumule donc des mesures nouvelles en dépenses, éminemment nécessaires, mais parfois insuffisantes, avec des propositions de baisse de prélèvements obligatoires, qui sont prises aujourd'hui à contretemps et qui pourraient, à tout le moins, être différées. Il s'agit, par exemple, de la suppression de la taxe d'habitation pour les 20 % de la population ayant les plus hauts revenus, pour 2,4 milliards d'euros cette année et 7,5 milliards d'euros annuellement au bout de trois ans. D'un côté, monsieur le ministre, vous souhaitez libérer l'épargne des gens qui en ont beaucoup, laquelle- vous l'avez dit, et cela a été chiffré -s'est beaucoup renforcée pendant le confinement, et, de l'autre, vous augmentez encore ces économies. Difficile à suivre Il en est de même de la baisse de l'impôt sur les sociétés, pour 3,7 milliards d'euros, qui s'ajoute aux réformes de la fiscalité du capital, dont le coût s'élève à 5 milliards d'euros par an et qui ont, elles aussi, bénéficié aux catégories sociales les plus aisées. Le Gouvernement fait également le choix de baisser les impôts dits « de production », pour un coût très important, de 10 milliards d'euros par an. Cette mesure, selon l'étude de l'Institut des politiques publiques, est ciblée non pas sur les entreprises fragilisées par la crise, mais plutôt sur les plus grosses, et beaucoup doutent de son efficacité. Le Gouvernement poursuit ainsi sa politique d'allégement de la fiscalité, sans prendre en considération son opportunité, alors que, dans le même temps, les dépenses publiques explosent. Par ailleurs, aucune mesure supplémentaire n'est prise pour mettre davantage à contribution, ne fût-ce que par un prélèvement exceptionnel, les entreprises qui sont les grandes gagnantes de la pandémie, Une crise de cette ampleur ne peut que se traduire par une augmentation de la dette. Pour autant, monsieur le ministre, vous ne faites rien pour en limiter le montant. Le commissaire européen

et qui seront confrontés d'ici peu à son remboursement constateront que vos décisions auront consisté à diminuer la participation des plus aisés, des actionnaires,

avait regretté, dès le mois de septembre 2019, l'abandon de toute velléité de programmation à moyen terme de nos finances publiques. À l'époque, le Gouvernement avait justifié cet abandon par les incertitudes entourant la réforme des retraites. Aujourd'hui, alors que la dette avoisine les 120 % du PIB, le ministre nous indique que la trajectoire et la situation de nos finances publiques nous obligent à une réflexion à moyen et long termes. De toute évidence, l'argument de la réforme des retraites a fait long feu ... On ne peut que regretter que cette réflexion, que chacun appelle de ses voeux, s'ouvre au plus mauvais moment, dans l'urgence d'une situation de crise économique et sanitaire. Je suis saisi,

Cette décision ne relève pas du rituel d'un opposant systématique. Elle n'est pas davantage une mesure dilatoire. Elle n'est pas non plus un imposé à l'ensemble des collègues, alors que des journées de débats intenses nous attendent dans cet hémicycle. Elle n'est rien de tout cela. Nous souhaitons proposer un moment pour essayer de prendre un peu de recul sur la situation économique, sociale et financière de notre pays. Les fins d'année relèvent toujours du marathon lors de l'examen du budget et nous laissent bien peu de temps pour mener des réflexions de fond. Cette tendance est renforcée par le présent exercice, compte tenu des conséquences lourdes de la pandémie, sur le plan économique bien sûr, mais aussi social. De ce point de vue, il y a urgence. urgence. Une question préalable, c'est aussi du temps de débat pour le Parlement, alors que le Sénat demande à être écouté et respecté par un exécutif qui tend trop souvent à enjamber le nécessaire débat parlementaire. Ce qui frappe, dans ce contexte inédit, c'est que les options fondamentales du Gouvernement ne sont nullement ébranlées par cette crise exceptionnelle. Vous vous entêtez ainsi, monsieur le ministre,

Cette réforme a accru la propension des ménages aisés à acquérir des titres en Bourse défiscalisés, sources de dividendes croissants sous-imposés. Un rapport récent confirme que les placements financiers des ménages les plus aisés sont passés de 45 milliards à 143 milliards d'euros entre 2017 et 2018. Les 1 500 premières fortunes de France ont chacune bénéficié d'une hausse des dividendes supérieure à 1 million d'euros. Vous comptiez sur le ruissellement. Nous en attendons encore les premières gouttes ! Vous nous expliquez que cette suppression a permis le retour en France d'exilés fiscaux. La différence entre les départs et les retours montre un solde positif de 77 personnes. Rappelons, à cet instant, que le nombre de foyers fiscaux assujettis à l'ISF, en son temps, était de 358 000. Vous n'avez pas mis fin au séparatisme fiscal Dans le même temps, nous pourrions évoquer la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, la, véritable bombe à retardement pour les finances publiques. L'écart de 15 points entre la taxation des salaires et celle des dividendes coûtera, à terme, 10 milliards d'euros par an, du fait des stratégies d'optimisation fiscale mises Trois années plus tard, il convient d'établir un état des lieux de la société française. Des rapports successifs mettent régulièrement en évidence l'aggravation spectaculaire des inégalités dans notre pays.

La France comptera, en cette fin d'année, 1 million de pauvres en plus, alors que le taux de pauvreté s'était déjà établi à 14,8 % de la population en 2018. De l'autre côté du spectre, la fortune des milliardaires français a augmenté de 439 % en dix ans, passant de 82 milliards de dollars en 2009 à 442 milliards en 2020, indépendamment du covid. La fracture sociale dénoncée un temps ne fait que s'aggraver. Banques alimentaires, Secours catholique, Secours populaire, Restos du coeur voient arriver dans leurs permanences des milliers de nouvelles familles. de solidarité active (RSA) dans les départements explose, parfois jusqu'à 40 %. Soyez bien conscients que l'urgence sociale est là ! Pandémie et confinement déstabilisent notre tissu commercial de proximité. Dans nos quartiers et nos communes, nous en faisons tous le constat. Pendant la même période, le e-commerce tire profit de la situation. La grande distribution, les compagnies d'assurances devraient contribuer fortement et davantage à la solidarité nationale.

Monsieur le ministre, vous refusez de taxer les hauts salaires et les dividendes et vous faites le choix d'avoir recours aux marchés financiers privés pour financer le budget. Ce faisant, vous choisissez la dette. Dans une réunion préparatoire de la commission des finances, notre rapporteur général, Jean-François Husson, faisait ce constat terrible, qu'il vient de rappeler : l'État français se finance désormais autant par l'endettement que par l'impôt. Nous nous retrouvons de plus en plus sous la tutelle de ces marchés financiers

l'État. La dette des États s'appelle « dette souveraine », mais on n'est pas souverain quand on dépend des marchés financiers ! Un pays est souverain quand le Parlement vote l'impôt, un impôt progressif, équitable et auquel, bien sûr, personne ne se soustrait.

Il nous faudra sortir du catastrophisme systématique, sans stigmatiser nos concitoyens qui seraient coupables de vivre au-dessus de leurs moyens et d'endetter leurs descendants, Dans l'Antiquité, on pouvait être condamné à l'esclavage pour dette. Il faudra bien sûr que l'État retrouve sa pleine souveraineté budgétaire, sa liberté, en imaginant d'autres moyens que le recours au marché privé pour assurer son financement. Non, l'État n'est pas le parasite proliférant au détriment de l'économie privée que l'on nous décrit si volontiers. S'il n'est pas seul à créer la croissance, il en est, du moins, l'un des paramètres essentiels. Depuis le printemps dernier, pas moins de 460 milliards d'euros d'aides en argent public ont été mobilisés sous diverses formes. Vous avez fait le choix de n'introduire aucun principe de conditionnalité à l'égard du monde économique, au nom de l'urgence, mais l'urgence n'est pas de revenir mécaniquement au monde d'avant. Cette crise bouscule, interroge. Le Président de la République, dans son intervention du 13 avril dernier, avait eu ces mots

Nous ne retrouvons pas ces belles envolées dans le projet de loi de finances qui nous est soumis : ce budget s'inscrit dans une continuité néolibérale qui ne répondra pas aux exigences de justice sociale. Le PLF se limite à la politique de l'offre et néglige fortement la demande. On n'y trouve rien sur les salaires, rien de significatif sur le pouvoir d'achat des ménages, si ce n'est quelques mesurettes, ici et là, sur la pauvreté. Franchement, le compte n'y est pas du tout. Une relance de l'offre dans un contexte de demande durablement anémiée, de gains de productivité inexistants, de taux historiquement faibles et de financiarisation n'a pas beaucoup de sens. Comment croire que ce budget est un budget de relance ? Les chiffres présentés sont sans ambiguïté : le volume des dépenses publiques recule sur un an. M. Le Maire s'est aussi félicité que le Gouvernement ne crée pas d'emplois publics. Or la pandémie a mis en évidence de manière très criante les immenses besoins dans nos hôpitaux publics, par exemple. En 2021, il y aura même une légère réduction nette d'emplois publics, avec 157 postes en moins. Certes, la communication autour des 100 milliards d'euros a été mais l'examen minutieux des dispositions budgétaires montre qu'il faut singulièrement nuancer ce chiffre. Quant aux 40 milliards d'euros de l'Union européenne, tout nous conduit à la plus grande prudence. Les 10 milliards d'euros de baisse des impôts de production viendront impacter fortement les budgets des collectivités bénéficiaires, alors que les collectivités ont elles aussi été en première ligne pour faire face à la pandémie ces derniers mois et restent encore, dans notre pays, un levier essentiel de la relance économique,

L'inquiétude quant à l'avenir grandit et la confiance recule. Oui, il faudrait demander un effort aux très hauts revenus. Il ne s'agit pas de punir qui que ce soit : il s'agit simplement d'essayer de construire des normes de justice acceptables pour le plus grand nombre.

Oui, il y a urgence à aller vers un système de plus grande justice fiscale. Ces débats ont lieu partout dans le monde. Il ne s'agit pas d'un tropisme français. Les mêmes questions se sont posées durant la campagne électorale américaine. Elles se posent au Royaume-Uni ou encore en Belgique. Telles sont, mes chers collègues, les raisons qui nous ont amenés à déposer cette question préalable.

monsieur le ministre, mes chers collègues, je serai d'autant plus bref que je suis absolument persuadé que, en leur for intérieur, nos collègues communistes n'ont absolument pas envie que nous votions cette question préalable.

nous avons des propositions à faire, car, une chose est certaine, le pays ne peut pas se permettre d'aborder l'année 2021 sans que nous votions des mesures fortes pour relancer l'activité. Je pense que nous pouvons tous être d'accord sur ce point. Le mieux que nous ayons à faire est donc de passer à la suite.

qui touchent aujourd'hui les commerçants, les indépendants, les petites entreprises. Le développement de ces acteurs, dans l'exercice de leur métier, et de leurs outils de production

tailles de conserver les emplois, aujourd'hui menacés à la fois par la crise et par la répétition des périodes de confinement. Enfin,

nous amène essentiellement à rembourser des intérêts et à renouveler le capital de la dette, d'où l'importance des taux d'intérêt, mais nous restons convaincus que la solvabilité et la crédibilité de l'État passent par son engagement et sa capacité à faire face à ses échéances et à rembourser. En cela, nous nous distinguons très nettement

les garanties d'emprunt et les prêts garantis par l'État, que vous avez inclus dans les dispositifs mobilisés pour faire face à la crise. En 2020, nous avons mis en oeuvre le Ségur de la santé, quelle que soit l'appréciation que vous pouvez porter à son sujet. nous avons franchi de nouvelles étapes en matière de mise en oeuvre du reste à charge zéro. Dès lors, je ne suis vraiment pas convaincu que le qualificatif « néolibéral » soit le plus approprié ! Je suis même convaincu du contraire.

je réaffirme ce que Bruno Le Maire a eu l'occasion de dire : nous avons besoin d'un peu plus de visibilité sur le rythme de sortie du confinement pour calibrer les mesures au mieux et faire en sorte que, nonobstant le risque d'un troisième confinement, que personne ne souhaite, le PLF pour 2021 puisse contenir les mesures nécessaires.

comme lui que le PLF est insuffisamment tourné vers les ménages, notamment vers ceux qui sont le plus en difficulté et qui basculent dans la pauvreté.

ce projet de loi de finances pour 2021 s'inscrit dans un contexte sanitaire, économique et social très compliqué- « exceptionnel », avez-vous dit, monsieur le ministre. Cette situation fragilise des pans entiers de notre économie et expose les plus vulnérables de nos concitoyens, elle met à mal les finances de notre pays et limite notre capacité à tracer les perspectives dont nous aurions pourtant besoin. Dans ce contexte inédit, le rôle de l'État est évidemment essentiel. Je le dis comme je le pense : l'État a été au rendez-vous pour maintenir le pays debout, grâce à un ensemble de mesures-

pour soutenir l'activité économique et l'emploi dans les territoires et pour organiser la solidarité dans la proximité, au plus près de nos concitoyens. Les collectivités territoriales constituent un point d'appui indispensable pour maintenir le pays en marche. C'est sur ce sujet des collectivités que je voudrais revenir à la lumière de cette première partie du projet de loi de finances ; mes collègues Sylvie Vermeillet et Vincent Delahaye évoqueront d'autres aspects de ce PLF. Avec les articles 3 et 4, vous proposez un allégement des impôts de production à hauteur de 10 milliards d'euros 7 milliards d'euros, par la suppression de la part régionale de CVAE, compensés par une part de TVA, et un peu plus de 3 milliards d'euros, avec la réforme des valeurs locatives des locaux industriels qui affecte le rendement de la compensés par un prélèvement sur ressources. C'est un pari pour favoriser la relocalisation de notre industrie et créer de nouveaux emplois, nos impôts de production étant deux fois plus élevés que la moyenne observée dans les pays de l'Union européenne. Toutefois, cette mesure affaiblit les recettes fiscales des collectivités et d'autres schémas seraient sans doute possibles- Sylvie Vermeillet reviendra Quoi qu'il en soit, nous devons veiller sans faiblir à la dynamique et à la pérennité des modalités de compensation aux collectivités locales. Ces dernières doivent garder leurs marges de manoeuvre, le pays en a besoin.

C'est un mécanisme pérenne et péréquateur alors qu'une compensation par une dotation de l'État, comme ce fut trop souvent le cas, reste aléatoire. Toutefois, la crise que nous traversons révèle une faille non pas sur le principe d'une compensation par la TVA, mais sur le mécanisme voté l'année dernière et sur lequel s'appuie la dynamique de cette recette : il n'est sécurisé ni pour les collectivités ni pour l'État. Nous comprenons donc la disposition prévue à l'article 22. Je le dis tranquillement : l'effet d'aubaine, ici favorable aux départements et défavorable à l'État, pourrait demain s'inverser. raison pour laquelle nous devons trouver une solution équilibrée et durable. Celle que vous proposez à l'article 22 apporte une réponse justifiée et juste, mais seulement pour 2022, pas au-delà. pas au-delà. Nous proposerons donc une autre solution afin de sécuriser durablement les recettes des collectivités et de l'État en cas de variation exceptionnelle des montants de la TVA perçue.

Nous proposerons également de corriger le traitement inéquitable entre les collectivités selon qu'elles subissent des pertes de recettes importantes, parce qu'elles gèrent leurs services et leurs équipements en régie,

Ne pensez-vous pas que nous devrions travailler à la mise en place d'un système lisible, stable, durable des ressources des collectivités locales ? Très bien ! Elles ont besoin de cette visibilité pour organiser le développement de leurs territoires. Dans l'attente, et nous reviendrons sur le sujet des collectivités lors de l'examen de la seconde partie de ce PLF, le groupe Union Centriste, dans sa très large majorité, adoptera la première partie de ce budget. Nous serons force de proposition pour enrichir le texte. Très bien

au Moyen Âge, d'intenter des procès aux animaux pour divers délits et crimes. C'est ainsi qu'à Autun, en pays bourguignon, au début du XVI siècle, un procès fut intenté aux rats de la ville l'on accusait d'avoir dévasté les récoltes de blé. Les paysans, en partie privés des fruits de leur travail, se trouvèrent dans l'incapacité de payer la dîme. Ils accusèrent alors les nuisibles. Après que justice fut rendue, on encouragea les paysans à se remettre au travail pour payer leur impôt. Depuis lors, les choses ont quelque peu changé. Quoique ... Il y a bien longtemps que l'on ne rend plus les rats, pas plus que les chauves-souris ou les pangolins, responsables de la diminution des ressources fiscales, et donc de la dégradation des finances publiques. Pourtant, en 2020, la tentation est grande de vouloir rendre un virus responsable de la situation catastrophique de nos finances publiques c'est à cause de la covid que notre pays affiche une récession à deux chiffres ; c'est à cause de la covid que le déficit dépasse les 220 milliards d'euros ; c'est à cause de la covid que notre taux d'endettement a bondi, en moins d'un an, de vingt points de PIB. Bref, c'est à cause d'un virus que nous nous apprêtons à examiner un budget historique pour la France, avec à la fois le déficit et la dette publics les plus élevés de notre histoire. La séquence budgétaire dans laquelle nous nous trouvons est sans précédent. Il est utile de nous le rappeler. Et il est utile, aussi, de nous rappeler que ce n'est pas le virus qui est responsable de cette situation catastrophique, mais bien les décisions que nous avons prises pour nous en protéger. Ce n'est malheureusement pas un scoop et ce projet de loi de finances pour 2021 s'inscrit dans la droite ligne des quatre projets de loi de finances rectificative pour 2020. Tous ces textes traduisent les décisions que nous avons prises collectivement pour lutter contre le virus. Ils correspondent au « quoi qu'il en coûte » que le Président de la République a lancé en mars dernier et qu'aucun responsable politique n'a réellement contesté. En clair, ils reflètent le choix que nous avons fait : donner la priorité à la santé des plus fragiles, quoi qu'il en coûte. C'est cette priorité donnée à la santé qui nous a collectivement conduits à ralentir le pays, à confiner les Français chez eux, à mettre nos entreprises sous cloche, à fermer les commerces. Et ces mesures radicales sans précédent ont converti la France entière, bon gré mal gré, à un néo-keynésianisme sous stéroïdes. Car tout découle de ces mesures radicales prises pour contenir la propagation du virus. Sans plan de sauvetage, nous aurions tué bon nombre de nos entreprises en 2020, la plupart dès le premier confinement et lors du second Aujourd'hui, sans plan de relance, nous laisserions notre économie exsangue face à la compétition mondiale : sans relance, impossible d'espérer renouer un jour avec la croissance ; sans croissance, impossible d'espérer rembourser les dettes astronomiques que nous avons contractées. C'est pourquoi, monsieur le ministre, nous avons à peu près accepté l'impérieuse nécessité d'engager de nouvelles dépenses sans augmenter les impôts. Face à la gravité de la situation, nous sommes nombreux à nous y résigner. D'autres exultent de voir enfin grand ouvertes les vannes de la dépense publique, et voudraient même ajouter de nouveaux impôts. Je n'entrerai pas dans le détail des différentes mesures dont nous aurons tout loisir de débattre au cours des trois prochaines semaines. je souhaite simplement présenter trois critères à l'aune desquels le groupe Les Indépendants examinera ce budget hors norme. Ces critères s'imposent à nous, alors que nous nous apprêtons à voter le pire déficit public de notre histoire. Le premier, c'est que ce budget de relance doit renforcer notre compétitivité. Il s'agit de nous assurer que chacune des mesures valorisera à la fois le travail et l'investissement, à la fois les efforts que feront les Français et les risques qu'ils prendront pour relever le pays. Ce n'est qu'à cette condition que nous sauverons le présent sans hypothéquer l'avenir. À cet égard, je tiens à saluer la baisse ambitieuse des impôts de production. Notre groupe l'appelait déjà de ses voeux lors du dernier projet de loi de finances. Ces impôts, parce qu'ils ne dépendent pas de la conjoncture, s'avèrent encore plus néfastes en temps de crise qu'en temps normal. Il était grand temps d'alléger ce fardeau qui obère la productivité des entreprises et pénalise l'économie de nos territoires face à la concurrence d'Europe et d'ailleurs. C'est pourquoi notre groupe soutient la baisse massive de la CVAE. Bien sûr, comme toute baisse des impôts, le risque existe, au moins à court terme, que certains y perdent. Nous serons donc particulièrement attentifs à ce que cette baisse ne se fasse pas aux dépens des collectivités locales, partenaires clés de la relance. Il y va de la cohésion de nos territoires, comme le soulignait à l'instant Bernard Delcros. Le second critère, c'est que la dépense publique contribue efficacement à préparer la France aux enjeux de demain. Le Gouvernement s'y est engagé. Nous y sommes aussi attachés. Notre groupe soutiendra les mesures qui favorisent l'investissement dans les technologies du futur et dans l'innovation partenariale, de même que les mesures qui facilitent la circulation des capitaux pour développer de nouvelles activités et celles qui encouragent la modernisation de notre outil de production. C'est dans le même esprit que notre groupe abordera les mesures visant à favoriser la transition écologique. Plus personne n'ignore l'urgence de la situation : « notre maison brûle », mais nous ne détournons plus le regard. La nécessité d'adapter nos modes de production et de consommation fait désormais consensus. À nous d'agir en conséquence. Il est urgent de protéger le climat et la biodiversité. Les priorités sont connues. Ainsi, nous devons faire preuve d'ambition pour lutter contre l'artificialisation des sols, pour réduire l'impact carbone de nos mobilités et pour améliorer l'efficacité énergétique de notre parc immobilier. Nous serons force de proposition pour renforcer le budget dans ce sens. Cependant, je veux être clair : nous ne chercherons pas pour autant à accéder systématiquement aux demandes de citoyens tirés au sort. L'enjeu est trop complexe, et surtout trop important, pour que nous nous contentions d'imposer et d'interdire pour engager la France dans une transition ambitieuse. Transition ne rime pas qu'avec taxation et restriction, comme le soutiennent les décroissants, mais surtout avec éducation et innovation. Nous ferons des propositions pour que la transition écologique soit adaptée à la réalité de nos territoires, à la ville comme à la campagne. Tous les Français veulent participer à cette transformation. Nous leur devons mieux que toujours plus de taxes et de contraintes.

Or pour ce faire, il n'y a pas d'échappatoire : il faut réduire au plus vite toutes les dépenses qui aggravent notre déficit structurel. La relance n'a de sens que si elle est temporaire, comme l'a rappelé le rapporteur général dans son L'objectif n'est pas de revenir à la situation que nous connaissions en 2019, mais bien de consolider la souveraineté de la France en renforçant la compétitivité économique et en accélérant la transition écologique. Mes chers collègues, « qui paie ses dettes s'enrichit » disait Balzac. Cela vaut tout autant pour notre dette publique que pour notre dette climatique. La parole

Au-delà des quatre plans d'urgence adoptés ici même depuis le début de la crise, le budget pour 2021 aurait dû être le moment clé de cette refondation, et ce d'autant plus qu'il s'agit du dernier budget en plein exercice du président Macron. Une refondation Et qu'observons-nous ? Une structure de budget inchangée par rapport à l'année dernière, assortie d'un plan de relance dont la majeure partie des crédits réellement opérationnels en 2021 ira à la réduction massive et sans contrepartie des impôts des entreprises. Tout sauf une refondation : une continuité, dangereuse. Où est la refondation quand on assiste à la poursuite de la baisse continue et massive de la fiscalité des entreprises ? ? Cette politique fiscale est une incessante course à la diminution des impôts des entreprises qui revient à faire reposer le poids de la dépense publique sur les ménages. Inefficace, elle exempte encore et toujours plus les grandes entreprises pourtant bien moins bien moins contributrices que les petites et moyennes entreprises et que les toutes petites entreprises dans notre pays. Et vous profitez de la crise pour aller encore plus loin. Nous reconnaissons bien là la « stratégie du choc », lorsque la sidération et la peur provoquées par la crise permettent de faire passer des mesures structurelles pour des mesures conjoncturelles. Voici ce que disait Guy Sorman en 1984, en observant, ravi, la politique de Ronald Reagan : « Le déficit engendré par la baisse des impôts apparaît comme un formidable moyen de pression pour contraindre l'État à rétrécir. » Quarante ans après, c'est ce que vous faites en faisant passer la baisse de 10 milliards d'euros par an d'impôts de production pour une mesure de relance. Mais derrière cette relance, par ailleurs surestimée, avec la baisse des recettes, c'est la bonne vieille méthode néolibérale : la création organisée de déficits qui servira, plus tard, à légitimer des mesures draconiennes afin de réduire à peau de chagrin les mécanismes de solidarité et d'ouvrir de nouveaux marchés à la sphère privée. C'est ainsi qu'il faut comprendre les propos de Bruno Le Maire dans les médias

Nous pouvons calculer tous les ans l'écart croissant entre l'accord de Paris, dont vous vous réclamez, et la réalité de l'action du Gouvernement. Je tiens à saluer l'action entreprise par Damien Carême, alors maire de Grande-Synthe, qui avait saisi le Conseil d'État pour « inaction climatique ». Cette dette s'accumule et nous ne pourrons négocier avec les banques pour la rembourser.

attendions alors à une diminution de la fiscalité des ménages après les demandes répétées et incessantes des Françaises et des Français pour rétablir les impôts des plus riches. Mais non On a surtout relevé, en guise de refondation, un entêtement à refuser toute forme de participation des plus riches à la crise. Avec obstination, ce gouvernement protège les riches. En ce domaine, il faut souligner banque UBS de juillet 2020 nous apprend que la France est classée au deuxième rang des pays pour l'augmentation du patrimoine des plus riches. Belle réussite ! le ministre. La République, invoquée tous les matins, n'est pas un glaive avec lequel on menace les citoyens. C'est d'abord un idéal de vivre ensemble où personne n'est laissé sur le carreau et qui devrait trouver une traduction concrète dans notre système d'imposition vous aviez là l'occasion de lutter contre le séparatisme fiscal qui fait ravage dans notre pays. Ce séparatisme des riches qui conduit la France à battre le record européen de versement des dividendes aux actionnaires dans une période de crise sanitaire où, nous le voyons tous dans nos territoires, la pauvreté explose. Où est la refondation quand vous refusez d'agir avec l'ambition nécessaire pour répondre au péril climatique ? que les lourdes exemptions fiscales accordées au monde économique ne sont conditionnées à aucune exigence de transition vers un modèle économique respectueux de l'environnement. Le Conseil d'analyse économique, rattaché à Matignon, montrait dans une note de juillet dernier que les trois premiers secteurs les plus favorisés par la baisse des impôts de production sont respectivement les producteurs d'électricité et de gaz, les industries extractives et la finance.

vous dotez la relance de l'économie verte de crédits nouveaux, mais vous fragilisez tous les instruments, à commencer par le ministère de l'environnement avec 770 postes en moins, qui doivent mettre en oeuvre ces politiques. Où est la refondation quand vous livrez à elles-mêmes les collectivités territoriales chargées de résoudre tous les problèmes des citoyens ? Le 13 avril dernier encore, le Président de la République disait aussi : « Au plus près du terrain,

Et pourtant, oui, nous avons besoin d'une refondation ! Pour cela, il aurait fallu un budget assorti d'une profonde réforme fiscale. Il aurait fallu un budget apportant un soutien bien plus important à l'économie sociale et solidaire, cette grande oubliée des plans de relance. Vous aviez l'occasion d'agir massivement pour cette économie au service des hommes et de la planète et vous ne faites que parer au plus urgent. Plutôt que de regarder, impuissants, les usines fermer, il faudrait un élan pour aider à la reprise par les salariés de leurs entreprises qui ferment, abandonnées par des actionnaires sans scrupules, pour la relocalisation et la fin de l'économie financiarisée. La refondation supposerait de prendre la mesure des transitions à venir. Vous prévoyez, par exemple, une aide aux entreprises pour leur transition numérique. Très bien, nous sommes d'accord, mais comment pouvez-vous ignorer les rapports et les études qui se multiplient et qui démontrent tous les jours un peu plus que les gains de productivité induits par la robotisation vont pousser à la disparition de très nombreux emplois peu qualifiés ? Les aides destinées à la numérisation des entreprises envisagées dans ce PLF ne sont pas accompagnées d'une vision ambitieuse pour permettre à la productivité ainsi dégagée de participer au financement de la protection sociale. Les mesures de formation ne seront pas non plus

Nous sommes dans une période où les transitions arrivent et la refondation n'est pas là. Ce budget ne refonde rien, alors que la situation que nous connaissons est en train d'aggraver toutes les crises que nous traversons. Monsieur le ministre, on n'invoque pas la République impunément, même si ce gouvernement le fait sans arrêt. Votre politique ne fait que la rendre plus abstraite, plus lointaine, parfois même plus hostile pour les Françaises et les Français qu'elle laisse sur le côté du chemin. Votre absence de vision d'avenir sur l'après-crise est dangereuse. Tout au long de l'examen de ce texte, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires essaiera de montrer les autres voies possibles. La refondation doit venir, nous sommes toutes et tous mobilisés pour essayer d'en chercher le chemin.

Quoi que l'on en dise, les chiffres sont et seront- hélas ! -toujours les chiffres. Nous avons beaucoup parlé de croissance et de récession, de dette, de taxes ou de dépenses, mais je souhaiterais que nous parlions ensemble de l'avenir. De ce qui fait, au fond, que nous soutiendrons ce budget et que nous préparerons ensemble l'après-crise pour nous et pour nos enfants. En effet, il serait vain de poursuivre cette longue litanie de chiffres qui occupe nos discussions depuis le début de l'après-midi sans donner un peu de perspectives. Nos concitoyens, nos proches, n'attendent pas telle enveloppe budgétaire ou telle mesure fiscale. Ils n'attendent pas non plus de savoir si le taux de croissance effectif rejoindra le taux de croissance potentiel. Ils attendent des réponses. Des réponses pour leur quotidien. L'assurance que l'État sera à leur côté

C'est ce qu'attendent nos voisins, nos amis, nos collègues, nos proches, de la Guyane à la Polynésie, en passant bien évidemment par l'Isère. Toutes celles et tous ceux qui se sont retrouvés du jour au lendemain en télétravail, ceux qui ont été confrontés à la fermeture de leur commerce, ceux d'entre nous qui ont été contraints de se tenir loin de leurs proches fragiles afin de les protéger, ceux enfin qui ont perdu un proche, un ami, un collègue et qui n'aspirent qu'à retrouver un peu d'humanité dans cette avalanche d'annonces dramatiques, de chiffres inquiétants et de mesures inhabituelles. C'est à ceux-là que je veux m'adresser aujourd'hui. À ceux pour lesquels nous renforçons notre soutien, budget après budget, texte après texte, à ceux qui attendent des réponses concrètes pour leur quotidien et qui s'inquiètent pour l'avenir et pour celui de leurs proches. À ceux-là mêmes qui ont été marqués par la crise que nous vivons et que nous tentons de traverser, chacun à notre manière. Vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, ils ont bénéficié de mesures de soutien courageuses cette année. Je pense notamment au financement du chômage partiel : nous sommes le seul pays au monde à avoir assuré le salaire de plus de 12 millions d'actifs. À situation exceptionnelle, budget exceptionnel. Alors que nos territoires sont frappés de plein fouet par la crise sanitaire, alors que les collectivités et les élus assument une nouvelle fois leurs responsabilités avec courage et opiniâtreté et accompagnent nos concitoyens face aux aux conséquences désastreuses auxquelles ils sont confrontés, qu'elles soient sociales ou économiques, alors que l'État confirme son soutien inédit aux entreprises, aux collectivités et à nos concitoyens, nous, parlementaires, devons être à la hauteur de leurs attentes. Nous le devons à ceux qui ont continué d'assurer leurs missions au plus fort de la crise. Nous le devons aux enseignants, aux soignants, aux éboueurs, aux ambulanciers, aux agents d'entretien, à tous ceux qui ont été en première ligne depuis le début de la crise. Mais nous le devons également à tous les agents des services de l'État qui n'ont jamais cessé de remplir leurs missions et qui ont déployé des trésors d'inventivité pour mettre en place des dispositifs de soutien, lesquels, reconnaissons-le, malgré une crise inédite qui a surpris jusqu'aux plus avisés d'entre nous, ont été d'une efficacité et d'une envergure sans précédent. C'est pour eux que nous devons examiner ce projet de loi de finances avec sérieux, rigueur et ambition. La crise actuelle nous oblige à réagir sans attendre et à déployer des moyens renforcés. Tel est l'objectif de la mission budgétaire spécialement abondée dans ce PLF pour alimenter le plan de relance. Ce dernier est indispensable pour atteindre les trois objectifs fixés par le Gouvernement, que sont le verdissement de l'économie, l'amélioration de la compétitivité des entreprises et le soutien aux plus fragiles. Ce plan de relance, ce sont 30 milliards d'euros alloués à la transition écologique, avec un plan ambitieux de rénovation énergétique et de transition agricole. Ce sont 34 milliards d'euros fléchés vers le soutien à la compétitivité et l'innovation, avec une nouvelle enveloppe de lutte contre la dépendance industrielle et technologique de notre économie et un plan de mise à niveau numérique des administrations et de nos entreprises. Ce sont, enfin, 36 milliards d'euros consacrés à la cohésion des territoires, avec un plan de modernisation du réseau routier ou de relance de l'activité dans les centres-villes. À quelque chose, malheur est bon, car les moyens nouveaux que nous devons déployer pour sauver notre économie seront au service d'une transformation profonde de notre économie, de nos infrastructures et de notre rapport à l'environnement. Ces trois priorités fortes et clairement assumées sont au coeur de ce plan de relance à 100 milliards d'euros, dont près de la moitié Seulement ? ... pour répondre au plus vite à l'urgence. Car l'urgence, c'est la relance, vous l'avez rappelé récemment, monsieur le ministre. Ces grands axes se traduisent par des mesures concrètes, dont certaines ont d'ores et déjà été inscrites au budget pour 2020. Dès la fin de l'année,

de faire cours à distance. Pensez donc à Valérie, professeure de français à Grenoble et personne à risque compte tenu de sa santé. Elle pourra continuer d'assurer l'enseignement de ses élèves à distance, grâce au recrutement d'un nouvel assistant d'éducation embauché dans son lycée. Cet effort sera sans aucun doute poursuivi dans ce budget pour 2021. Le PLF pour 2021, c'est un budget qui accompagne également la rénovation énergétique des bâtiments, avec la transformation du crédit d'impôt pour la transition énergétique en une aide, « MaPrimeRénov' », alimentée d'un budget considérable de 2 milliards d'euros pour la seule année 2021. Pour Jean, jeune entrepreneur et propriétaire d'une maison, l'État prendra en charge le quart de ses dépenses de rénovation thermique. Avec ce budget, les entreprises pourront aussi réaliser des travaux de rénovation énergétique. Pour son entreprise, Jean pourra bénéficier d'un crédit d'impôt accessible pour les dépenses engagées depuis depuis le 1 octobre et prenant en charge 30 % des travaux entrepris. Pour Jean, le PLF pour 2021, c'est également une baisse inédite des impôts de production,

qui financera à hauteur de 5 000 euros l'envoi en mission d'un VIE par son entreprise. L'État finance avec toutes ces mesures un plan de relance d'une ampleur inédite, il n'oublie pas pour autant de soutenir les plus démunis. Car la précarité guette bon nombre de nos concitoyens, parmi les populations les plus fragiles et les plus atteintes par la crise. Elle menace notamment les jeunes de notre pays, étudiants comme jeunes diplômés. Dans le PLF pour 2021, le Gouvernement confirme sa volonté de s'attaquer à la question de la précarité, en renforçant le dispositif garantie jeunes et en facilitant les nouvelles aides à l'embauche. C'est également l'une des raisons pour lesquelles notre groupe soutiendra ce projet de loi de finances. Alexandre, lui, est un jeune boursier de 20 ans à l'université. On sait qu'il est difficile d'avoir 20 ans en 2020. Pourtant,

qui pourra s'ajouter à ses revenus d'activité, dans le cadre de la garantie jeunes. Pour Alexandre, l'État propose également une aide exceptionnelle créée dès la troisième loi de finances rectificative, d'un montant de 4 000 euros par an, qui permettra à une entreprise de l'embaucher en CDI ou CDD de trois mois et plus, pour un salaire jusqu'à deux fois le SMIC. S'il cherche à être embauché dans le cadre d'un contrat d'alternance, le PLF pour 2021 le soutiendra également, en accordant à l'entreprise un montant pouvant aller jusqu'à 8 000 euros. Mais

Ce PLF s'inscrit dans la continuité des actions que nous menons résolument depuis trois ans en faveur des territoires. Il s'agit de redonner du pouvoir aux élus locaux et de les replacer au coeur des territoires, avec la loi Engagement et proximité, de favoriser la revitalisation des territoires, avec les programmes Action coeur de ville, Petites villes de demain et Territoires d'industrie, d'accélérer la transition écologique par le biais des contrats de transition écologique ou le déploiement des mobilités durables. durables. Au coeur de la crise sanitaire, l'État n'a pas failli et a accompagné les collectivités, notamment par les mesures d'urgence prises dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative, à l'origine de la mise en place du « filet de sécurité budgétaire » pour les collectivités du bloc communal. dispositif de soutien ambitieux permet de compenser les pertes de recettes engendrées par la crise sanitaire et économique. Le dispositif d'avances remboursables des DMTO permet également de préserver les finances des départements. Le PLF pour 2021 comprend des mesures fortes d'accompagnement des collectivités locales dans la relance économique. D'une part, il prévoit le maintien historique des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales pour 2021, avec une dotation globale de fonctionnement à hauteur de 26,8 milliards d'euros,

le PLF prévoit la compensation intégrale et dynamique de la baisse des impôts de production. La CVAE régionale sera intégralement compensée par une fraction de TVA affectée aux régions. Les communes et les EPCI bénéficient d'une compensation dynamique et territorialisée de l'allégement de la fiscalité sur les établissements industriels, un nouveau prélèvement sur les recettes de l'État, à hauteur de 3,3 milliards d'euros.

Enfin, vous le savez, ce PLF pour 2021 sera marqué par l'entrée en vigueur de l'acte II de la suppression de la taxe d'habitation, votée dans le cadre de la loi de finances de l'an dernier. Le PLF pour 2021 constitue donc un engagement inédit, à la hauteur de l'accompagnement attendu par les collectivités, qui se poursuit dans le cadre du plan de relance, dont 1,5 milliard d'euros bénéficieront directement aux territoires ultramarins. Le groupe RDPI soutient les bases du projet de loi de finances pour 2021. Solidaires de l'action du Gouvernement, mais vigilants s'agissant de la mise en oeuvre de la relance, nous proposerons

En mars dernier, il a fallu préserver la santé de nos concitoyens. C'était nécessaire, mais nous ressentons aujourd'hui les conséquences de ce choix, même si nous ne pouvons encore en mesurer toute l'ampleur, d'un point de vue non

Des mesures budgétaires ont aussitôt été prises pour financer l'urgence sanitaire et compenser les pertes brutales de revenus et de chiffre d'affaires. Beaucoup a été fait lors de la première vague. Malheureusement, nombre de nos compatriotes, les plus fragiles, sont cruellement atteints par ce deuxième confinement et se demandent s'ils pourront en surmonter le coût. Afin d'en contrecarrer les effets, le projet de loi de finances pour 2021 s'inscrit dans la continuité des mesures d'urgence entérinées par les quatre projets de loi de finances rectificative successifs, sans oublier le plan de relance, inscrit dans le budget général pour 2021 comme une mission à part entière, pour un montant de 36,4 milliards d'euros en autorisations d'engagement. Alors que la sortie du premier confinement durant l'été avait apporté une dynamique de reprise et que les analyses prospectives présentées en commission des finances laissaient entrevoir un rétablissement budgétaire, le deuxième épisode de confinement nous oblige à revoir à la baisse nos hypothèses de rebond. La pandémie est venue bouleverser intégralement toutes les prévisions, et la discussion budgétaire en porte les stigmates. La situation économique et financière de notre pays s'est dégradée avec cette crise sanitaire, mais la loi de finances pour 2021, si elle répond à l'urgence et à la situation conjoncturelle, n'amorce aucun changement de direction par rapport à la situation de l'avant-crise. Les crédits des missions les plus significatifs restent ceux de la mission « Enseignement scolaire », avec 54,9 milliards d'euros, soit une progression de 1,4 milliard d'euros, de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », pour 26 milliards

le rappelle, les projets de loi d'urgence sanitaire ont permis de pallier les conséquences sociales de la crise sanitaire, même si le coût de la dette qui en découle demeure une inquiétude. Ainsi, le remboursement des 10 milliards d'euros apportés par l'Union européenne dès 2021 pourrait représenter des annuités de l'ordre de 2,5 milliards d'euros à compter de 2028. Mais revenons aux mesures budgétaires en tant que telles. La baisse annoncée de 10 milliards d'euros des impôts de production des entreprises est maintenue, avec pour objectif affiché la souveraineté et la relocalisation des emplois industriels. l'article 3 prévoit la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et un ajustement de la contribution économique territoriale (CET) pour cet impôt qui s'élève, en France, à 77 milliards d'euros, soit le double de la moyenne de L'article supprime la part régionale de la CVAE, qui représente 50 % du total, et lui substitue une fraction supplémentaire de TVA. Le plafond de la CET passe de 3 % à 2 %. Avec moi, les membres du groupe du RDSE regrettent qu'aucune réelle contrepartie sociale ou écologique ne soit exigée. Nous redoutons que cette mesure ne favorise les grandes entreprises, alors que ce sont véritablement les plus petites d'entre elles qui sont en danger, car elles sont davantage pénalisées par le deuxième confinement. Elles représentent pourtant un gisement d'emplois non délocalisables, précieux pour maintenir la vie et le lien social au coeur de nos territoires. Déjà, de très nombreux artisans, commerçants ou prestataires de services estiment qu'ils ne seront pas en mesure de rembourser les prêts garantis par l'État. Leur survie est compromise, à l'image du secteur de la culture, du tourisme, des loisirs, des festivals, de la restauration, des services à la personne, pour ne citer que ces quelques exemples.

Malgré les 4 milliards d'euros consacrés à l'entrée dans la vie professionnelle des jeunes et les 5 milliards d'euros prévus pour le volet « cohésion » centré sur la sauvegarde de l'emploi, le chômage partiel ou la formation, nous craignons que les plus fragiles ne paient le prix fort des conséquences de ce deuxième confinement. Autre lacune de ce budget pour 2021, l'insuffisance des moyens octroyés aux collectivités territoriales non seulement pour faire face aux surcoûts consécutifs à la gestion de la crise sanitaire, mais aussi pour tenir une place prépondérante dans la relance économique. Au travers des aides et de la reprise des investissements, elles auraient pu jouer un rôle moteur, un rôle de levier, pour contribuer à la relance économique, en assurant le maintien des investissements et de la commande publique. La loi de finances ne tient pas ses promesses en la matière, et le compte n'y est pas pour les collectivités territoriales

L'article 3 prévoit l'élargissement du champ de la déduction pour épargne de précaution aux aquaculteurs et aux centres équestres, autant de mesures qui seront utiles concrètement, tout comme celles qui sont prises en faveur des entreprises du secteur du théâtre ou du spectacle,

C'est une évidence, la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2021 se caractérise principalement par une très forte inquiétude. Selon les différentes hypothèses retenues concernant la situation sanitaire ou encore la durée ou la sévérité du confinement effectif, les prévisions de croissance varient et restent fragiles. La prévision de solde effectif est de-6,7 % du PIB,

La perte d'activité de novembre serait moindre que celle du printemps : 12 % au lieu de 30 % en avril. Selon les données de la Banque de France, elle serait plus modérée

Dans ces conditions, le déficit public devrait atteindre 11,3 % du PIB, pour un endettement de 119,8 %. Nous devons tabler sur des prévisions de croissance prudentes à l'issue du reconfinement. En conclusion, nous pouvons affirmer que, pour 2021, l'État se finance autant par l'endettement que par l'impôt. Mais chacun le sait bien ici, les emprunts d'aujourd'hui sont les impôts de demain. Conscient que notre pays s'inscrit dans un effort financier somme toute plus faible que celui déployé par certains de nos voisins européens, le groupe du RDSE sera très soucieux, au cours de la discussion budgétaire, de maintenir la dynamique de nos territoires et la solidarité envers les plus fragiles de nos concitoyens, dans un souci d'équité. La parole

Monsieur le président,

le Président de la République et le Gouvernement ont souvent rappelé que nous étions en guerre contre le virus. Cette métaphore guerrière est dangereuse pour la démocratie et l'unité du peuple, à l'image du précédent couvre-feu, décision d'exception qui a une histoire dans la société française. Je vous le dis, monsieur le ministre, les mots ont toujours des conséquences La crise sanitaire fait des ravages économiques et sociaux. Les économies qui ont été confrontées à de tels chocs se sont toujours reposées sur trois piliers nationalisation et planification des secteurs fondamentaux, taxation des bénéfices exceptionnels liés à la crise et mise en place d'un circuit de financement des dépenses publiques, indépendamment du marché. Ces choix politiques ont été pris au sortir d'événements historiques douloureux, ne l'oublions pas. L'histoire n'est pas sans leçons. Alors que l'observation de la conjoncture est une exhortation à changer de cap, vous vous contentez de reconduire la même politique de l'offre, selon une conditionnalité relative dans l'octroi de l'argent public, et c'est peu dire : elle est très forte pour les plus précaires, mais pratiquement absente pour les grandes entreprises. Cette approche déconnectée de la réalité a favorisé le coup d'éclat de la droite, samedi dernier, sur l'âge de la retraite, confortant ainsi l'insécurité sociale. Cette loi de finances pour 2021 doit être l'ébauche d'une nouvelle vision politique, celle d'une redistribution la plus juste et la plus équitable, celle qui répond aux vrais besoins. Nous, sénatrices et sénateurs du groupe CRCE,

Il y a bien, dans cette loi de finances, des mesures d'urgence, mais l'urgence sociale vous échappe. C'est le budget de l'état actuel du capitalisme, où prédominent la technocratie et le marché. Monsieur le ministre, vous avez dit à mon collègue Éric Bocquet que vous ne meniez pas une politique néolibérale. Vous n'êtes pas néolibéral, vous n'êtes pas ordolibéral, vous n'êtes pas ultralibéral ... Mais qu'est-ce que vous êtes libéral, monsieur le ministre ! Que dire des méthodes ? dire des méthodes ? Sans m'alarmer sur les inquiétantes questions de la réduction du temps de débat public ou de la dépossession du Parlement de ses pouvoirs de vote de l'impôt et de contrôle, que penser de l'absence de concertation entre acteurs et bénéficiaires de ce budget ? Votre conception de l'État trouve ses sources dans une forme de surdité politique entretenue. Elle constitue le fil rouge de vos politiques d'après-crise, pour défendre une forme illusoire d'« autorégulation naturelle » des injustices criantes. La surdité aux aspirations populaires au changement porte déjà votre signature, et vous persistez pourtant à vous enfoncer dans une continuité aveugle, qui n'a rien de « disruptif

Notre groupe propose de transformer un texte de loi suscitant lassitude et défiance en un budget d'émancipation humaine et démocratique. Nous voulons traiter les urgences de la vie des Françaises et des Français ; nous voulons ouvrir un horizon plus juste et plus égalitaire. L'audace exigerait d'abord de rééquilibrer le rapport entre le travail et le capital. Le travail productif engendre directement une plus-value économique et une valeur sociale. Il est réalisé par les travailleurs : je pense aux infirmières, aux livreurs, aux ouvriers, aux personnels d'entretien ... À ce sujet, j'écoutais ce matin à la radio Patrice Blanc, président des Restos du coeur,

Nous sommes aujourd'hui face à des personnes effectuant des activités essentielles, qui, si elles décidaient demain d'arrêter de travailler, provoqueraient l'effondrement d'un système économique qui s'est reposé sur leur sous-rémunération et leur exploitation. Il est grand temps que cela cesse Comment accepter que les 20 % les plus riches voient leurs richesses croître énormément pendant et après le confinement, quand les 20 % les plus pauvres continuent de plonger dans l'endettement et la misère ? Grâce au travail improductif, la rémunération du capital a engendré toujours plus de richesses pour ceux qui en détiennent : les 10 % des Français les plus riches ont amassé plus de la moitié des 32 milliards d'euros de surcroît d'épargne accumulée pendant la crise. La réponse doit être simple et directe, à savoir une taxation exceptionnelle des revenus ayant bénéficié aux foyers les plus riches et aux entreprises dont les profits ont explosé. L'audace exigerait également d'arrêter de vouloir réduire massivement les dépenses publiques au profit d'une succession de privatisations de services, qui, aujourd'hui, nous font défaut. Je pense notamment aux secteurs de l'énergie des transports ferroviaires, mais aussi à l'hôpital public et à la recherche. Nous sommes confrontés à une marchandisation qui traite spontanément des biens sociaux comme des biens privés. Parlez-leur de maillage du territoire et de petites lignes, on vous répondra indicateur de rentabilité d'une rame ou fréquence de passagers. Si l'État doit intervenir, ce n'est pas pour enrichir les actionnaires ni pour se rendre complice des suppressions d'emplois ou d'une détérioration du climat. Pas d'aides publiques pour les entreprises qui trichent ! Je pense tout particulièrement aux Gafam, objet de notre amendement déposé lundi dans le cadre du PLFR 4 et visant à la création de la notion d'établissement stable. J'ai d'ailleurs bien noté le double langage tenu dans certaines travées de cet hémicycle, qui consiste à soutenir l'amendement en séance, mais à le retoquer en CMP. Ce n'est pas la première fois ! Parler des services publics pose la question des services d'intérêt général et des choix démocratiques. Relocalisons l'économie et évitons les drames sociaux chez Goodyear, Bridgestone, Carrefour, et d'autres. Ayons du cran ! Ne faisons pas croire que les réponses à la crise sont trop complexes, ce sont avant tout des choix politiques. Mes chers collègues, notre État de droit est devenu un État de la faveur, où tout se monétise, y compris notre souveraineté. Puisque nous parlerons d'emprunt, quelles réponses structurelles trouve-t-on dans le budget proposé pour contrer l'aggravation de la dette privée, qui s'élève à 150 % du PIB au second semestre de 2020 ? L'encours de la dette des entreprises privées a doublé. Enfin, comment pouvez-vous fermer les yeux sur l'absence de taxation des transactions financières ? transactions non essentielles bénéficient pourtant d'un passe-droit de TVA, contrairement à d'autres biens de première nécessité. Nous ne lâcherons pas sur ces sujets. La continuité budgétaire se manifeste aussi à l'égard des collectivités. La démocratie locale est menacée par la perte d'autonomie fiscale.

assistons à la disparition des impôts locaux, remplacés par des dotations liées au produit des impôts nationaux. Chaque année, la marge de manoeuvre des élus locaux se réduit, et l'autonomie fiscale des collectivités n'aura d'autonomie que le nom. Cette hypercentralisation des budgets locaux doit cesser ! Elle est tout le contraire d'une démocratie vivante ! La position du Gouvernement est une faute démocratique et politique. En faisant disparaître la responsabilité fiscale et, donc, politique des assemblées locales élues au suffrage universel, c'est le fondement même de la démocratie qui est sapé. Le consentement à l'impôt comme moyen de financer les charges communes crée une responsabilité des élus, mais également des citoyens et des entreprises. Sans cela, la démocratie locale perd tout son sens.

et 3 millions d'actifs. Pourtant, on n'en parle pas ! L'intelligence du local, que possèdent nos élus grâce à leur expérience et la connaissance de leur collectivité et de leur population, est essentielle. À l'heure du deuxième confinement, le constat est sans appel les finances locales subissent des pertes de plusieurs milliards d'euros. Le cercle de l'endettement devient insoutenable pour les collectivités, qui, privées de leurs marges de manoeuvre budgétaires, ne pourront pas participer à la relance. En effet, la commande publique est en baisse de 22 % par rapport à 2019. Les départements voient leurs dépenses sociales alourdies par la précarisation de la population. Les collectivités locales sont fragilisées, et vous ne répondez au principal que par de l'accessoire. Nous répondrons par des amendements visant à les sécuriser financièrement. Mes chers collègues, « le bonheur existe et j'y crois » disait Aragon aux heures sombres.

2021. Ce que nous savons déjà, en revanche, c'est que la crise a fait basculer 1 million de nos concitoyens dans la pauvreté, en plus des 9 millions qui étaient déjà dans cette situation. La Fondation Abbé Pierre a rappelé a rappelé récemment que près de 300 000 personnes sont aujourd'hui sans domicile fixe dans notre pays, soit deux fois plus qu'il y a dix ans. Dans ces circonstances exceptionnelles, l'enjeu principal de ce budget est donc le plan de relance

il faut bien sûr ajouter la baisse de 10 milliards d'euros des impôts de production. Cette réduction d'impôts sur les entreprises nous interroge elle n'est soumise à aucune contrepartie ou presque, que ce soit en matière d'emploi, de responsabilité sociale des entreprises ou de transition écologique. S'agissant d'un tel montant- vous en conviendrez, monsieur le ministre -, c'est un pari risqué. Cette action, qui porte sur l'offre et se veut structurelle, reste, quoi qu'on en pense, une réponse décalée face à une situation conjoncturelle aussi grave et exceptionnelle que celle que nous vivons. Elle ne résoudra pas à elle seule la brutale récession économique que nous traversons. Des économistes ont proposé d'autres solutions ; ainsi, celle français des conjonctures économiques : « Plutôt que de baisser les impôts de production, il aurait mieux valu annuler les dettes des entreprises liées au covid-19, comme les charges sociales C'est pourquoi, avec le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, entre autres mesures pour plus de justice fiscale, mais aussi pour plus d'efficacité dans la promotion d'un nouveau modèle de développement à l'issue de cette crise, nous proposerons de revenir sur cette baisse des impôts de production ou d'exiger au moins leur conditionnalité. Nous proposerons le rétablissement de la tranche supérieure de la taxe sur les salaires pour les entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA sur la totalité de leur chiffre d'affaires nous proposerons également la suppression ou l'atténuation de la « niche Copé », dispositif d'optimisation fiscale, ainsi qu'un changement des modalités de calcul du crédit d'impôt recherche, afin d'en encadrer l'utilisation par les grands groupes. Nous proposerons par un élargissement de la taxe sur les surfaces commerciales aux activités de stockage de type Amazon, et la hausse de la taxe GAFA. Nous en parlons depuis si longtemps ; avançons enfin ! Dans la même logique, et afin de venir en aide aux commerçants qui sont particulièrement touchés par la crise au bénéfice des géants du numérique, nous proposerons une contribution exceptionnelle des grandes surfaces et des acteurs du e-commerce pour alimenter un fonds de soutien aux commerces de proximité. En refusant obstinément de faire contribuer ceux qui le peuvent, et même ceux qui profitent de cette période de crise, le Gouvernement se prive de moyens pour agir en faveur des victimes de la crise et, en même temps, fait le choix du déficit public. Le niveau de la dette publique devrait par conséquent atteindre, à la fin de l'année 2020, 120 % du PIB ; elle n'est soutenable que grâce au niveau toujours plus bas des taux d'intérêt.

Pour lutter contre l'aggravation des inégalités sociales, nous pensons qu'il faut changer d'approche ; la crise le nécessite encore davantage. Vous avez déjà été contraints de faire ce changement d'approche, certes très modestement, dans dans le budget pour 2019, à la suite de la crise des « gilets jaunes ». Lors de l'examen du dernier projet de loi de finances rectificative, au début de la semaine, vous avez refusé nos propositions en ce sens, au motif qu'elles seraient examinées lors de la discussion du projet de loi de finances. Il est temps N'attendez pas une nouvelle explosion sociale. Notre pays a besoin de justice fiscale ; la période exige d'aider davantage les victimes de la crise et de faire participer davantage les plus fortunés à l'effort de solidarité nationale. Ainsi proposerons-nous la réinstauration d'un impôt sur le capital pour remplacer l'ISF et la suppression de la. Nous proposerons aussi de relever le plafond des dons au profit des associations d'aide aux personnes en difficulté. Parce qu'il n'est pas normal que notre pays laisse tant de jeunes sans perspectives et surtout sans moyens, nous proposerons la création d'une dotation « autonomie jeunesse Destinée aux 18-25 ans, elle leur permettrait de disposer des ressources auxquelles ils n'ont plus accès en raison des restrictions actuelles d'activité. La présidente du Secours catholique Véronique Fayet le disait ce matin sur France Inter- nous sommes nombreux à l'avoir entendue - : « Dans cette situation de crise, il faut que les jeunes aient un accompagnement renforcé [ ...], mais avec cela il faut qu'ils soient soutenus par une allocation digne. de la discussion du projet de loi de finances rectificative, lundi dernier, la majorité sénatoriale a rejeté, main dans la main avec le Gouvernement, tous nos amendements destinés à lutter contre la pauvreté.

? Il faut passer d'une prise de conscience et des paroles aux actes ; la discussion budgétaire nous en donne justement l'occasion. Les autres grands oubliés de ce budget sont bien sûr les collectivités locales. La baisse des impôts de production est pour elles une nouvelle perte d'autonomie fiscale.

chers collègues, ce PLF apparaît très imparfait et fort déséquilibré : oubli de la jeunesse, réponse incomplète à la crise, hausse des déficits sans perspective de retour à l'équilibre, nouvelle fragilisation des collectivités locales.

qui « marche » dans la situation que nous vivons. Pourtant, nous sommes aujourd'hui face au dernier « vrai » budget du quinquennat. Avons-nous devant nous un budget de relance, comme le dit le Gouvernement,

dans ce plan de relance, qui vise pourtant à toucher tout le monde, des oubliés, notamment les plus démunis- cela a déjà été dit à plusieurs reprises. L'augmentation générale des minima sociaux, réclamée sur certaines travées, nous s'inscrire dans un vrai débat sur la redistribution et l'architecture de nos prélèvements et transferts destinés aux plus précaires. Nous soutiendrons, dans le cadre de ce texte, des mesures exceptionnelles et temporaires, pour favoriser l'emploi des jeunes Je note aussi une absence de mesures d'économies structurelles, visant certainement à ne pas déplaire. Les crédits des missions baissent facialement ... pour mieux se retrouver dans le plan de relance. Le groupe Les Républicains n'a pas peur de dire qu'il va falloir collectivement faire des efforts.

Cette relance que vous nous annoncez, nous considérons qu'elle débute avec six mois de retard. En juillet, notre groupe avait déjà proposé un certain nombre de mesures ; 90 % des dispositions présentées par le Gouvernement n'entreront en vigueur qu'en 2021 ou en 2022 ! C'est beaucoup trop tard ; l'Allemagne, par exemple, a commencé bien avant nous. Certaines Certaines des mesures que vous nous avez refusées en juillet ont été reprises par le Gouvernement en septembre. Je citerai, entre autres, la baisse des impôts de production, les mesures en faveur des jeunes et de l'apprentissage, ou encore l'extension de la prime remplaçant le crédit d'impôt Je relève donc avec malice que nous n'avons pas toujours de mauvaises idées ! Nous soutiendrons bien évidemment l'ensemble des dispositifs qui visent à baisser les impôts de production. Il n'est question en la matière, malheureusement, que d'une goutte d'eau : même en comptant ces mesures, nous resterons encore très loin de l'Allemagne et des autres pays de l'Union européenne.

C'est le temps de la dépense publique. » Un de ses prédécesseurs avait pourtant eu le courage de dire, en avril 1998, à l'Assemblée nationale : « Il nous faut abandonner l'idée qu'en matière de dépenses publiques, " plus " est synonyme de " mieux " . » Vous aurez tous reconnu là les propos de Laurent Fabius Nous croyons qu'il vaut mieux sacrifier des recettes fiscales de demain et limiter l'endettement d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous vous proposerons des mesures de déblocage de l'épargne forcée des ménages en faveur d'un soutien aux fonds propres des entreprises. Le surcroît d'épargne des ménages atteindra 100 milliards d'euros à la fin de l'année, soit le montant de votre plan de relance. Nous pensons également que les collectivités territoriales doivent être au coeur de cette relance- je vous rappelle qu'elles représentent plus de 70 % de l'investissement public. C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons notamment un versement contemporain des Par ailleurs, depuis deux ans, votre gouvernement nous annonce un. Malheureusement, j'ai plutôt l'impression d'être face à un budget vert J'ai lu le « jaune » budgétaire : seuls 10 % des 574 milliards d'euros de dépenses du PLF pour 2021 sont considérés comme ayant un impact sur l'environnement. Nous sommes très loin des déclarations que faisait Bruno Le Maire au mois de septembre : « Grâce à ce budget vert, nous présentons l'impact environnemental de tous les crédits budgétaires et de toutes les dépenses fiscales de l'État. » Nous n'avons certainement pas la même définition du mot « toutes » Nous pourrons vraiment parler d'un budget vert lorsque le PLF se caractérisera par une augmentation significative des crédits en faveur de l'écologie. En tant que rapporteur spécial, je fais un constat simple : à périmètre constant, les crédits consacrés à l'écologie, à l'environnement et à la mobilité durable baissent de 6 %. Nous pourrions améliorer la démarche en réservant une partie du débat budgétaire à l'évaluation climatique des lois de finances et en organisant un suivi de cette évaluation par un organe spécialisé, sur le modèle de la Mecss, la mission d'évaluation et Je pense d'ailleurs qu'il serait intéressant de procéder à une évaluation du coût de la tonne de CO2 évitée par les mesures du plan de relance. Les premiers chiffres qui circulent l'évaluent à plusieurs centaines d'euros Le groupe Les Républicains souhaite une écologie moins punitive. Nous proposerons notamment- nous suivrons M. le rapporteur général -le lissage sur cinq ans de la hausse du malus. Je note d'ailleurs que, en la matière, vous revenez sur votre parole. Certaines décisions peuvent paraître incompréhensibles ; par exemple, comment allez-vous prendre en compte le bilan carbone d'une voiture moins lourde, mais fabriquée en Chine ? Comment allez-vous prendre en compte les situations particulières où l'achat d'un véhicule de plus grande taille empêche la circulation de plusieurs véhicules de plus petite taille ? Nous voterons également pour la suppression du malus sur le poids, qui, vu toutes les mesures d'exception que vous proposez, ne concernera que 1 % du parc- reconnaissez que nous sommes là face à une mesure démagogique, qui aura pour seule conséquence de fragiliser notre industrie automobile. Si encore l'ensemble des recettes du malus étaient affectées à la transition écologique ... Que nenni ! Il ne s'agit que d'une mesure de rendement budgétaire. Nous voulons surtout plus d'écologie positive. Très bien ! Nous proposerons une hausse des crédits de la prime à la conversion, un encouragement au télétravail et un déblocage anticipé de l'épargne salariale pour l'achat d'un véhicule propre ou la réalisation de travaux de rénovation thermique. Il nous semble également que l'accès à l'excellence environnementale ne doit pas être ouvert uniquement aux plus aisés. Je donnerai deux exemples. Pour un foyer dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur à 13 489 euros, le montant maximal d'aide publique pour l'achat d'un véhicule électrique est de 12 000 euros.

Par ailleurs, l'incitation à la rénovation thermique reste faible pour les propriétaires bailleurs, car elle est fortement conditionnée, notamment par un encadrement des loyers. Et ce ne sont pas eux qui paient ensuite les factures de chauffage des logements Ce budget, vous l'aurez compris, ne nous rassure pas et ne donne pas confiance dans l'avenir. Les contribuables s'effraient de l'envolée de la dette de l'État et de la dette sociale ; ils savent qu'il faudra bien les rembourser. Ils s'attendent tôt ou tard à voir leurs impôts augmenter- j'ai bien noté que Bruno Le Maire s'était engagé à ce que tel ne soit pas

qui pourront demain faire partie des variables d'ajustement. La parole de l'État, elle, est sans cesse remise en cause. Je citerai trois exemples tirés de ce seul projet de loi de finances : la remise en cause des dispositions votées l'année dernière quant à la compensation de la perte des recettes

Contrairement à ce que le Gouvernement indiquait dans le cadre du débat d'orientation des finances publiques, nous n'avons pas aujourd'hui un « budget de relance et de souveraineté au service des priorités écologiques et sociales Nous n'avons pas un budget qui donne confiance dans l'avenir. Rien ne sera possible, pourtant, sans un changement de comportement des consommateurs, qui doivent être incités à dépenser l'épargne de précaution qu'ils ont accumulée depuis plusieurs mois. Tant que les Français n'auront pas confiance dans la reprise de l'économie, l'épargne forcée du premier confinement continuera à se transformer durablement en une épargne de précaution. Nous vous le disons : sans confiance, pas de croissance

le traditionnel examen du projet de loi de finances prend cette année une dimension exceptionnelle. Il s'établit dans un contexte profondément marqué par la crise du coronavirus. L'instabilité sanitaire est devenue budgétaire. À titre personnel, je sais qu'il ne pouvait en être autrement, sauf à laisser notre santé publique, notre économie, nos emplois et notre modèle social sombrer. Dans le prolongement des quatre lois de finances rectificatives de l'année écoulée, et afin de répondre à l'impact économique et social de la crise sanitaire, ce PLF est un projet de relance et d'espoir. Fondé sur une hypothèse de croissance de 8 % en 2021, il est censé s'inscrire dans un temps de rebond économique. Il reste que financer la relance par la croissance ne sera pas chose aisée.

notre ministre de l'économie et des finances, qui déclarait devant nos collègues députés, cet été, que « les impôts de production sont de mauvais impôts, des impôts stupides, parce qu'ils pèsent sur les entreprises avant même qu'elles aient fait des bénéfices Cependant, en l'état, le texte cible exclusivement les impôts économiques locaux et réduit une nouvelle fois l'autonomie fiscale des collectivités territoriales. Au nom du groupe Union Centriste, je défendrai un amendement visant à atteindre la bonne cible en supprimant la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) dont sont redevables les entreprises qui réalisent plus de 19 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Ce faisant, l'État et les collectivités partageraient l'abandon d'un impôt : 4 milliards d'euros pour l'État sans C3S et 4,6 milliards d'euros nets pour les collectivités sans CFE et sans CVAE.

Le Sénat doit porter leur message, leurs inquiétudes. Il doit proposer tout ce qui préservera le dynamisme et la volonté des territoires. Nous avons une solution : partager l'effort, c'est-à-dire supprimer l'impôt local pour les petites structures, qui sauront apprécier l'allégement consenti, et supprimer la C3S pour les grandes qui, de toute façon, viendront réclamer cette suppression. Tôt ou tard, et même après la disparition de l'impôt local, les grandes entreprises nous expliqueront de nouveau combien la C3S est nocive pour leur compétitivité, combien elle est exclusivement française, donc illégitime. Si nos fleurons nationaux gagnent en compétitivité, l'État sera l'autre grand bénéficiaire. d'analyse économique estime que la suppression de la C3S permettrait de réduire le déficit de la balance commerciale de plus de 5 milliards d'euros. Telle est aussi l'hypothèse du groupe Union Centriste, et nous en débattrons. Mais n'oublions pas que l'État a tout autant besoin de collectivités fortes que d'entreprises fortes. Elles savent d'ailleurs très bien grandir ensemble. Laissons-les vivre en synergie ! La parole

nous voilà donc à l'examen du projet de budget pour 2021. Que constatons-nous ? Nous constatons que, en quelques mois, toutes les doctrines budgétaires ont volé en éclat toutes les règles de limitation des dépenses publiques sont devenues obsolètes ; tous les verrous et carcans d'hier, qu'ils soient nationaux ou communautaires, ont sauté. Sous nos yeux et au gré des PLFR successifs, ce qui était jusqu'alors impossible est advenu, et même devenu vital. En termes comptables, nous convenons naturellement que l'effort budgétaire consenti cette année et celui prévu pour l'an prochain sont très importants. Toutes les missions ou presque voient leurs crédits augmenter, et le plan de relance semble enfin s'engager. Cet effort, ce déficit et cet endettement, l'Europe les comprend, la Cour des comptes les comprend, chacun de nous ici les comprend et, par endroits, les approuve. Mais, si nous les comprenons, souffrez aussi que nous émettions des doutes sur l'exécution de ce budget et sur la répartition de l'effort, donc sur son efficacité.

comment croire en effet que, au-delà des milliards annoncés, les crédits inscrits seront bel et bien consommés ? L'expérience vécue outre-mer nous apprend en effet à être méfiants. Mes chers collègues, le budget d'une nation est bien plus qu'une addition arithmétique de milliards. Un budget, c'est un acte politique, la traduction d'une philosophie, d'une vision, année après année, de l'avenir d'une société. Or, par-delà les montants exceptionnels qui sont présentés, ce que nous contestons fondamentalement dans ce budget, c'est bel et bien son orientation

dont le bourgeois aime à peupler son monde à lui, le meilleur des mondes possibles », et ce parce qu'elle ne parvient pas ou renonce même à « pénétrer l'ensemble réel et intime des rapports de production dans la société. » Vous aurez trouvé de quel auteur il s'agit ... La philosophie que nous mettons en cause est bien celle du libéralisme à tous crins, du monétarisme et de l'inégalitarisme cette croyance fétichiste dans la supériorité du marché qui est celle de l'individualisme possessif et gourmand. Cette crise a mis à l'épreuve votre cette crise était donc pour vous l'occasion de changer de paradigme et de trouver, en quelque sorte, sorte, votre chemin de Damas. Cette théologie du salut individualiste souffre d'une déficience épistémique dont, j'en suis sûr, vous avez parfaitement conscience. Mais, malgré les démentis infligés à vos choix économiques et sociaux, vous persistez dans cette politique darwiniste qui centralise, qui fragilise, qui précarise. Regardez la partie relative aux recettes : aucun effort demandé aux plus fortunés ; rien sur la fiscalité patrimoniale ou successorale ; rien pour faire face à la voracité des multinationales ; rien pour soutenir l'épargne populaire- je déposerai des amendements en ce sens ; si peu pour soulager nos collectivités locales

Bruxelles la critique. La soutenabilité financière des collectivités est donc de nouveau menacée ; leur autonomie fiscale est une fois encore mise à mal. Bien que la dureté de la réalité sociale vous rattrape, vous restez figés et arc-boutés. Votre surmoi libéral est plus fort que la réalité des faits. Les faits, c'est une augmentation de 9 % du nombre de bénéficiaires du RSA prévue l'an prochain ; les faits, c'est, sur le terrain, des associations de lutte contre la précarité en plein désarroi depuis la fin des contrats aidés ; les faits, c'est un marché du travail tellement précarisé depuis trois ans qu'il insécurise même ceux qui garderont leur emploi ; les faits, c'est l'spéculative et prédatrice des sociétés d'investissement, qui échappent toujours à toute réglementation. Non, vous ne partez pas de nulle part ; depuis 2017, votre politique est mue par l'idée selon laquelle les inégalités créent la croissance et les vices privés font la vertu publique, raison pour laquelle vous avez continuellement abaissé la fiscalité sur les plus riches ; raison pour laquelle vous avez continuellement privilégié les libertés économiques des plus forts aux solidarités sociales pourtant nécessaires.

Et ce ne sont pas les 700 millions d'euros annoncés au forceps et fin octobre qui changeront la donne. C'est purement indigent ! Nous sommes des parlementaires responsables. Nous sommes même des parlementaires inventifs et combatifs, qui persistons à vous démontrer que d'autres voies sont encore possibles. Parce que cette crise touche d'abord les plus précaires, nous vous proposerons, au cours des débats, une véritable boîte à outils, exposée plus tôt par notre collègue Rémi Féraud. Parce que nous croyons encore à la belle phrase dite par Lacordaire en 1844 : « Entre le faible et le fort, entre le pauvre et le riche, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui affranchit. » Nous le voyons, votre utopie libérale et individualiste s'est muée en dystopie sociale. Quel sera donc votre legs ? Derrière ces milliards, fictifs ou tangibles, la question qui nous obsédera dès l'an prochain et pour cinquante ans encore est celle-ci : qui paiera en dernier ressort l'explosion de la dette ainsi créée ? Nous vivons un impensé de la dette et restons dans l'orthodoxie la plus indigente. On prend avec condescendance l'idée de dettes perpétuelles ou de très long terme, ou celle d'une possible suppression des dettes souveraines. Le dogme de l'orthodoxie monétaire et bancaire étouffe et aveugle. Vous évitez ainsi d'ouvrir tout débat relatif à un possible effacement partiel de la dette pour préserver, dites-vous, la crédibilité de la signature française. Cette inclination persistante est, je vous le dis, proprement irréaliste et idéologique. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, à l'aube de ce débat, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ne désespère pas de corriger les biais inégalitaires, darwiniens et kafkaïens de ce PLF. Bon travail à tous

sur la forme comme sur le fond, sur le conjoncturel comme sur le structurel, sur l'économique comme sur le social, pour aujourd'hui et pour demain

un programme regroupe les crédits destinés à mettre en oeuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère ». Force est de constater que votre mission « Plan de relance » et ses programmes ne répondent pas à cette exigence de la LOLF

Alors, il y a l'investissement, mais vous le savez comme moi, monsieur le ministre, toutes les entreprises aujourd'hui bloquent leurs investissements. Les collectivités, qui ont des ressources en moins, ont elles aussi arrêté d'investir. Tout cela constitue un risque majeur. La consommation repartira, mais uniquement si vous rouvrez les commerces

! Je ne critique pas les lois de finances rectificatives : nous les avons votées pour vous aider, monsieur le ministre, pour aider le Gouvernement et pour aider la France. En revanche, je n'estime pas que le « quoi qu'il en coûte » et la valse des milliards, qui constituent dorénavant l'unité de compte du budget, soient de bons indicateurs pour les réformes à venir. La dette, je l'ai entendu, sera remboursée par la croissance.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, 520 milliards d'euros de dettes nouvelles en deux ans ! On finance tout à crédit ! Ces 520 milliards sont à comparer aux 100 milliards d'euros consacrés au soutien et à la relance : cela fait quand même réfléchir Certes, ce budget ne finance pas que du soutien et de la relance. C'est la valse des milliards, on est en pleine dérive budgétaire, on augmente les effectifs, on augmente les rémunérations des fonctionnaires. trois exemples symptomatiques parmi d'autres. Premier exemple, 425 créations d'emplois sont prévues pour les agences régionales de santé. On renforce l'administration du système de santé alors que l'on devrait transférer des moyens de l'administration vers le médical et les soignants. Deuxième exemple, plus de 10 milliards d'euros seront consacrés aux ministères, contre zéro euro pour les collectivités ! La loi de finances renforce le pouvoir central au détriment des territoires. Troisième exemple, les effectifs du Conseil d'État et de la Cour des comptes sont renforcés, et avec eux le pouvoir des juges. Parallèlement, le pouvoir des élus est encore affaibli en raison d'une nouvelle diminution de leur autonomie fiscale.

On vient de célébrer les cinquante ans de la mort du général de Gaulle, cet homme d'État dont le courage n'était pas la moindre des qualités. Rappelons-nous que, en 1958, à la demande du général, le plan Pinay-Rueff prévoyait, pour revenir à l'équilibre du budget, une baisse de 14 % des dépenses publiques. Quel courage ! Résultat : envolée de la croissance pendant dix ans Notre gestion absurde de la crise, selon, qui rebaptise la France « Absurdistan », nous coûte cher, très cher

merci aux Chinois, à l'Arabie Saoudite, mais surtout aux banques centrales et à l'Union européenne, sans lesquels nous ne pourrions plus fonctionner aujourd'hui

l'économie : pour rembourser la dette, il faut de la croissance, il faut une gestion saine des finances publiques et il faut des réformes structurelles. Mais dans la réalité, c'est autre chose.

économie. J'aimerais que l'on me prouve que la croissance future est compatible avec les objectifs très ambitieux que nous nous sommes fixés en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

dire des réformes structurelles, troisième pilier du remboursement souhaitable de notre dette, sinon que c'est l'Arlésienne dont on parle toujours et que l'on ne voit jamais venir ? La gestion catastrophique du projet de réforme des retraites en est un triste exemple. Mes chers collègues, notre réaction à l'épidémie et les faiblesses de notre système de santé nous ont mis à plat budgétairement, économiquement et socialement. Tout est lié. Mais la crise a bon dos ! Sous couvert de crise, on amplifie la pratique du laisser-aller budgétaire. Les Français sont anesthésiés par la peur, mais aussi par les milliards qui pleuvent. Attention, monsieur le ministre, le réveil sera brutal et douloureux À titre personnel, sans doute avec quelques collègues ayant toujours été attachés à une gestion rigoureuse de l'argent public, je voterai contre ce projet de loi de finances. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, face à la crise sanitaire, désormais également sociale et économique, qui ronge notre pays, ce projet de loi de finances pour 2021 était attendu, de permettre la relance de toutes les forces de la Nation et de redonner du souffle aux Français. Le compte n'y est malheureusement pas, mais les mécomptes y sont Combien de chiffres alarmants, monsieur le ministre, combien de rapports soulignant les effets inadaptés de vos mesures vous faudra-t-il encore pour changer de cap ? Nous sommes face à un PLF sans grande surprise, dans la droite ou devrais-je plutôt dire dans la ligne de droite ? -d'une politique libérale plus ou moins assumée ! Vous faites preuve d'une confiance inébranlable dans la main invisible du marché et dans la politique de l'offre pour régler les problèmes, entre habituels cadeaux aux multinationales et aux plus riches, et renoncement à une vraie solidarité. solidarité. Le Gouvernement fait clairement le choix de poursuivre la réduction des impôts pour les grandes entreprises et les ménages les plus riches, alors même que les besoins en recettes seront essentiels pour renforcer les services publics et rembourser les dettes engendrées par la crise du coronavirus. Le Gouvernement parie encore sur la croissance alors que celle-ci est affaiblie et qu'elle peinera à rebondir, conformément à ce que l'on constate depuis plus de cinquante ans. C'est un fait établi que vous devez prendre en compte dans vos prévisions. Il va falloir de nouveau questionner notre définition de la croissance : il y a urgence à le faire Dans un contexte où la croissance ne reviendra pas au niveau espéré, il nous faut trouver les moyens de satisfaire les besoins des Français de manière juste et équitable. Vous n'en prenez pas le chemin dans ce projet de budget Quelle stratégie guide votre nouvelle baisse massive des impôts pour les entreprises ? Pour quelle compétitivité et pour quels emplois prenez-vous de telles décisions ? C'est une politique qui essuie pourtant des échecs évidents. Je pense à Air France et à Renault, qui ont reçu des aides en début d'année et envisagent aujourd'hui des licenciements. J'aurais pu également citer Engie, Airbus et bien d'autres. Comment ne pas évoquer l'absence ou l'insuffisance de contreparties exigées pour ces entreprises dans le domaine social ou environnemental ?

C'est ce que l'on peut appeler le ruissellement à l'envers ! Toujours en matière de stratégie, je suis très étonné que l'on trouve dans la mission « Plan de relance » le programme 362, « Écologie », qui n'a rien à y faire. Tout d'abord parce qu'il ne produira que des effets limités en 2021 et surtout parce que la transition écologique est nécessairement un processus de long terme. Dès lors, il doit s'agir d'une mission structurante et non conjoncturelle. Avant même un plan de relance, il aurait d'abord fallu un plan de soutien, car la crise sanitaire ne va pas se terminer le 31 décembre de cette année. Un plan de soutien est nécessaire pour les entreprises qui sont au bord de la faillite. Je pense, en particulier, aux restaurants, aux bars, aux cafés, aux petits commerces et à bien d'autres, qui risquent de ne pas bénéficier du plan de relance tout simplement parce qu'ils n'existeront plus.

Ces derniers mois, le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire a augmenté d'environ 30 %, voire de plus de 45 % dans certains départements. Où sont les crédits ouverts au bon niveau pour les plus démunis dans ce PLF ? À côté d'une politique de soutien que nous appelons de nos voeux, vous l'aurez compris, l'efficacité d'une véritable relance doit passer par les territoires, tous les territoires, en particulier par ceux que je connais le mieux, à savoir les territoires ruraux, en nous appuyant notamment sur les collectivités locales.

Cette année, en raison de la pandémie, les collectivités locales devraient enregistrer des pertes financières nettes de l'ordre de 3 milliards d'euros, en l'absence de compensation suffisante de la part de l'État. À cela s'ajoute le mécanisme de bascule des impôts de production, prélevés sur les entreprises au niveau local, vers des impôts sur la consommation prélevés, notamment sur les ménages, au niveau national. Les collectivités territoriales perdent ainsi la main sur une part importante de leurs recettes, qui leur garantissaient

PLF manque d'une stratégie renouvelée sur l'évolution à long terme de la société française que cette crise impose. Pour demain, quel tournant écologique, quel plein emploi, quelle souveraineté alimentaire, quelle souveraineté industrielle, quelle souveraineté technologique, quelles justices fiscale et sociale ? Autant de réponses à ces questions que nous ne percevons pas ! La parole

Bien évidemment, cela ne signifie pas que le niveau du déficit budgétaire et de la dette publique nous soit soudainement devenu indifférent. Si l'on ajoute aux

Jusqu'à présent, grâce à la baisse des taux devenus même négatifs, à la politique de la BCE et à la gestion de France Trésor l'emballement de notre dette a été indolore, mais 2020 sera la dernière année où son coût diminuera alors même que le stock enfle : ce sera terminé Il est donc temps, monsieur le ministre, de mettre en place une stratégie de désendettement, qui passera probablement par le cantonnement de la dette dite « covid » et l'affectation d'une ressource pérenne

! Pour l'heure, quatre questions nous sont posées, et je ne doute pas qu'elles structureront nos débats. Faut-il, dès 2021, alourdir la fiscalité des particuliers ou des entreprises pour dégager des moyens supplémentaires, comme certains le demandent ? Ce n'est pas le choix du Gouvernement, et je pense qu'il a raison. Les mesures de soutien à nos entreprises en difficulté sont-elles bien ciblées et suffisantes ? Je crois que le débat n'a pas été clos par le PLFR 4. Même question pour les mesures de relance de ce PLF- j'y reviendrai. Enfin, dernière question, et pas la moindre, les aides aux Français les plus touchés par cette crise empêcheront-elles un basculement massif et durable des plus précaires dans la pauvreté ? Malheureusement, la tendance est inquiétante. Que ferons-nous ?

Les mois perdus, combinés aux effets du reconfinement, risquent de rendre inatteignable l'objectif, affiché par Bruno Le Maire il y a quelques semaines seulement, d'un effacement des effets de cette crise sur notre PIB dès 2022. Pour espérer tenir cet objectif ambitieux, il nous faudrait réunir plusieurs conditions. faudrait préserver notre potentiel de croissance et donc soutenir massivement nos entreprises, grandes ou petites. De gros efforts ont été réalisés en ce sens, nul ne peut le nier, mais chacun voit bien venir le moment où, malgré les reports de charges, le fonds de soutien, le PGE et le dispositif beaucoup de PME ne tiendront pas en cas de prolongement du reconfinement ou si un troisième confinement s'avérait nécessaire, dans l'attente d'un vaccin. Il nous faut donc, dès maintenant, réfléchir à cette hypothèse et agir. dire à tous ces chefs d'entreprise, artisans et commerçants, qui ne savent pas s'ils pourront passer la fin de l'année, ce que le Gouvernement entend faire pour eux. Il nous faut ensuite un plan de relance massif et ciblé sur les secteurs susceptibles de redémarrer rapidement, malgré la crise sanitaire. Nous le savons, notre pays est pénalisé par la structure même de son économie, où des secteurs comme le tourisme et l'aéronautique pèsent lourd. Ceux-ci ne retrouveront pas leur niveau d'avant la crise avant plusieurs années. Nous devons donc, d'un côté, soutenir plus longtemps et plus fortement ceux qui devront attendre la reprise et, de l'autre, investir massivement dans les secteurs où la demande intérieure est le principal moteur. C'est le cas du logement, monsieur le ministre, point que je développerai à présent. Car la construction neuve est bien l'angle mort de ce plan de relance, comme elle est en réalité l'angle mort de votre politique depuis 2017. Pourtant, les besoins sont immenses au-dessous de 500 000 logements neufs par an, nous ne répondons pas aux besoins, et le décalage entre l'offre et la demande qui s'accroît fait continuellement monter les prix, aggravant par là même la crise. Or qu'avez-vous fait depuis trois ans ?

suppression de l'APL accession, économies sur les aides fiscales avec le resserrement du prêt à taux zéro (PTZ) et du Pinel. Ajoutez à cette liste le resserrement du crédit bancaire et vous avez l'explication de ce qui est en train de se passer

Monsieur le ministre, j'évoquais le besoin de visibilité des acteurs économiques. Quand dissiperez-vous le brouillard qui entoure également les acteurs du logement ? Entendons-nous bien. Rechercher la plus grande efficacité de la dépense publique : nous sommes d'accord. Trouver des économies : ce pays va devoir le faire. Mais la question est bien de savoir où et avec quelles conséquences ! Depuis trois ans, vous nous répétez que vos réformes permettront un « Élan » nouveau pour la construction, selon le titre de la dernière loi. Résultat : en 2020, on financera moins de 100 000 logements sociaux et, pour la première fois, tous types de logements confondus, le nombre des autorisations de construire accordées sera inférieur au nombre des mises en chantier. Les courbes se sont croisées : le pire est devant nous nous ! Reconnaissez au moins que vous vous êtes trompé et changez de stratégie ! Si la mode est au Grenelle, il en faut un sur le logement, auquel il faudra associer étroitement les élus locaux. Car tout se tient et la disparition de la taxe d'habitation, comme la non-compensation des exonérations de taxe sur le foncier bâti,

Souvenez-vous-en, monsieur le ministre, particulièrement en cette période de crise et acceptez, dès ce PLF, un certain nombre des amendements que nous allons vous proposer sur le sujet. La parole

Le PLF pour 2021 était donc l'occasion pour le Gouvernement de traduire cette volonté d'un acte II du quinquennat orienté vers la proximité et les collectivités territoriales.

En tant qu'ancien maire de Houssen et président de l'association des maires du Haut-Rhin, département le plus touché lors de la première vague de covid-19, j'ai pu voir le dévouement de mes collègues sur le terrain. Partout dans le pays, les élus locaux ont été au rendez-vous en maintenant les services publics essentiels et en palliant les défaillances de l'État, au-delà du champ habituel de leurs compétences.

5 milliards du plan France Relance fléchés vers les collectivités ; maintien des dotations, notamment de la DGF ; augmentation de la DSIL à un niveau historiquement haut ; majoration de la dotation générale de décentralisation pour les régions

La suppression de la TH pour le bloc communal et celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les départements pourraient avoir des conséquences importantes en matière de potentiel fiscal et de péréquation.

Pour les communes, la taxe d'habitation est remplacée par le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur lequel s'appliquent un coefficient correcteur et un abondement de l'État prélevé sur les frais de gestion sur la fiscalité locale. En matière de simplification, on a vu mieux ! Pour comprendre le mécanisme de la baisse des impôts de production, c'est encore pire. C'est un processus de transferts, de compensations fractionnées, de plafonnements, de revalorisations des valeurs locatives, etc. C'est encore plus compliqué et alambiqué. Je ne sais pas s'il y a des plombiers à Bercy, mais c'est une belle tuyauterie qui nous est proposée : un véritable centre Pompidou de la fiscalité

Les départements vont subir un véritable effet ciseaux entre l'augmentation du RSA et la diminution de leurs recettes. Pour le département du Haut-Rhin, on observe déjà une augmentation de 12,5 % du nombre de bénéficiaires du RSA à l'issue de la première vague, ce qui représente un coût supplémentaire de 10 millions d'euros pour la collectivité. Les intercommunalités et les communes font face à un risque avec les pertes de recettes liées à l'activité. C'est dans cette optique que le rapporteur général présentera un amendement tendant à compenser la perte de recettes en 2021 pour le bloc communal et pour le bloc départemental.

Chaque euro versé a un effet multiplicateur. Monsieur le ministre, mes chers collègues, au-delà de ces éléments, c'est surtout une nouvelle approche et une nouvelle relation entre État et collectivités qu'il convient d'impulser dans nos territoires. Le grand débat national avait déjà posé le constat ; la crise sanitaire, puis économique l'a confirmé. Pourtant, nous voyons encore surgir les vieux réflexes des excès de centralisation et d'un fonctionnement trop vertical. Par exemple, lorsqu'il s'agit de territorialiser le plan de relance, l'État met en place des sous-préfets dédiés à la relance, alors qu'il suffirait de faire confiance aux forces vives des territoires ! Cette gestion digne de « l'ancien monde » ne peut pas répondre efficacement à l'attente de nos concitoyens. Désormais, il convient d'enclencher une véritable logique partenariale entre l'État et les collectivités. Libérons les énergies sur nos territoires ; laissons les collectivités prendre des initiatives et innover ; capitalisons sur le couple maire-préfet, qui commence à montrer son efficacité

pertinente. L'État doit désormais se poser en accompagnateur et en facilitateur dans sa relation avec les collectivités. Car la proximité est aussi l'affaire de l'État, qui doit améliorer la présence de ses services sur le terrain. Je pense notamment aux maisons France Service dans les cantons. Monsieur le Monsieur le ministre, mes chers collègues, vous l'aurez compris, le PLF pour 2021 aurait dû marquer un changement de philosophie à l'égard des collectivités. Ce n'est malheureusement pas encore le cas.

Au Sénat, chambre des territoires, nous y serons évidemment très attentifs et nous serons force de propositions, sur le fondement notamment des cinquante mesures de plein exercice des libertés locales présentées au mois de juillet dernier par le président Gérard Larcher et par MM. Philippe Bas et Jean-Marie Bockel.

que toutes les dépenses de transfert ou de salaire ne seraient pas évaluées au regard de leur effet sur l'environnement, considérant que c'était par principe neutre. Nous sommes évidemment ouverts à une évolution méthodologique sur ces points. Il est important de le noter, nous avons procédé à cette évaluation tant sur

l'engagement et la traçabilité des efforts des entreprises dans le domaine de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que pour le dialogue social et la consultation,

est plus viable, plus simple et plus pérenne. Le fait de compenser par une fraction de TVA ou par un prélèvement sur recettes avec une indexation sur les valeurs locatives a le mérite à la fois de la simplicité et du dynamisme. Quatrièmement-

Effectivement, l'État fait le choix de financer ses priorités et de garantir le maintien des dotations qu'il verse aux collectivités locales. Reprocher au Gouvernement d'augmenter les crédits des ministères plutôt que les dotations aux collectivités n'est pas compatible- je le dis comme je le pense

le fait que cette mission relève, pour sa programmation et son exécution, du seul ministère de l'économie, des finances et de la relance. C'est un choix politique de pilotage du plan de relance. J'assume également- je l'ai dit dans mon intervention liminaire et devant la commission des finances -, le fait de n'avoir construit que trois programmes,

pour la deuxième partie, ce qui nous permettrait d'avoir un fléchage précis ? Je ne comprends pas qu'il faille chaque fois

Si je devais en faire une démonstration, je me référerais aux débats que nous avons eus sur le PLFSS. C'est au Sénat que nous avons actualisé l'article liminaire. C'est également au Sénat que nous avons proposé d'adopter des dispositions complétant les crédits en matière de dépenses hospitalières, de dépenses de santé et d'objectif national

Monsieur le ministre,

ayant été déposés sur cette première partie -, nous vous proposerions d'actualiser de nouveau l'article liminaire en tenant compte de l'effet de la nouvelle prévision tant sur les recettes que sur le niveau du déficit.

relatif à la participation de la France au budget de l'Union européenne. Au préalable, il est nécessaire de rappeler que notre contribution dépend directement de l'issue des négociations du prochain cadre financier pluriannuel (CFP). Après deux ans de négociations houleuses, les États membres ont trouvé un accord sur le budget pluriannuel de l'Union européenne lors du Conseil européen qui s'est tenu du 17 juillet au 21 juillet dernier. Cet accord a été obtenu dans un contexte de fortes attentes des citoyens européens sur la réponse à apporter à la crise. Dans cette perspective, l'accord de juillet constitue un tournant budgétaire et politique majeur. Il définit un CFP dit « socle », s'élevant à 1 074 milliards d'euros en crédits d'engagement, complété par un instrument de relance de 750 milliards d'euros. Le Parlement européen a négocié une hausse de 16 milliards d'euros du CFP. Cette somme qui devrait être ciblée sur les éléments jugés prioritaires par le Parlement européen, comme Erasmus ou les L'articulation entre le CFP socle et cet instrument de relance retient un schéma inédit, avec, pour le second, un financement assuré par des ressources levées sur les marchés financiers par la Commission européenne, au nom de l'ensemble des États membres. Toutefois, la commission des finances estime que des interrogations subsistent sur la mise en oeuvre du nouveau CFP et du plan de relance. La première, et non des moindres, tient au veto opposé par la Hongrie et la Pologne, rejointes hier par la Slovénie, sur le mécanisme de conditionnalité des fonds européens. Il met en péril l'adoption pour le 1 janvier du nouveau CFP et du plan de relance européen.

depuis le début des négociations en 2018, le Sénat n'a eu de cesse d'alerter sur les risques d'un éventuel retard de celles-ci, retard qui serait très préjudiciable pour les porteurs de projets locaux, en particulier dans le domaine de la politique de cohésion. Cette crainte devient aujourd'hui une véritable angoisse, alors que le calendrier paraît plus contraint que jamais. Un déblocage de la situation vous semble-t-il possible dans les prochaines semaines ? Quelles seront les conséquences d'un échec sur le projet de budget pour 2021, première année du nouveau CFP ? deuxième interrogation concerne la gouvernance et le décaissement des crédits de la facilité. La procédure de décaissement est guidée par le souci de garantir que les sommes issues de l'endettement de l'endettement commun sont utilisées à bon escient, mais force est de constater qu'elle est complexe et longue. Dans ces conditions, il paraît évident que les plans de relance nationaux restent en première ligne pour assurer le soutien à la reprise économique. Il faut être transparent : le plan de relance européen constitue bien un remboursement des dépenses engagées par les États membres dans leur plan de relance national. La commission des finances a exprimé des inquiétudes quant au coût du plan de relance pour la France. En effet, en l'absence de nouvelles ressources propres, le remboursement sera assuré par les États membres en fonction de part dans le revenu national brut de l'Union européenne. Pour la France, le remboursement du plan de relance européen pourrait s'élever à 2,5 milliards d'euros par an. Certes, le Conseil européen a fait de l'introduction de nouvelles ressources propres une priorité. Toutefois, la tâche reste immense pour aplanir les désaccords entre les États membres en la matière. Alors que le Parlement européen estime que le calendrier de la mise en place de nouvelles ressources propres est « juridiquement contraignant », le Conseil considère qu'il s'agit d'une simple feuille de route, témoignant ainsi du caractère sensible du sujet. En tout état de cause, il faudra être particulièrement vigilant pour que ces nouvelles ressources propres ne soient pas vécues comme la création d'un impôt supplémentaire par nos concitoyens.

une part significative de la hausse de ce montant s'explique par le retrait du Royaume-Uni du budget européen. Mais il convient de rappeler que l'accord du mois de juillet dernier a modifié les règles de calcul des contributions nationales. Cela se traduit par un ressaut de 700 millions d'euros pour la France en 2021. À cet égard, l'accord de juillet a entériné un renoncement de la France sur la question des rabais. Si le coût budgétaire aurait pu être mieux maîtrisé, il est certain que le coût politique d'une absence d'accord aurait été beaucoup plus élevé. En outre, la France a tout de même réussi à faire prévaloir certaines de ses positions sur le plan des dépenses, notamment en matière de politique agricole commune. Sous réserve de ces différentes observations, je recommande, au nom de la commission des finances, d'adopter sans modification l'article 31 du projet de loi de finances pour 2021. La

31 matérialise la participation de la France au budget de l'Union européenne pour la première année du nouveau cadre financier pluriannuel, un CFP en discussion depuis le mois de mai 2018, et je sais de quoi je parle ... Ce nouveau CFP, complété par un instrument de relance en réponse à la crise de la covid-19, devait marquer une nouvelle étape pour l'Union européenne, une étape de solidarité, dont l'emprunt réalisé au nom de l'Union européenne est la marque symbolique. Ce paquet budgétaire venait de faire l'objet d'un accord entre la présidence allemande du Conseil européen et le Parlement européen, qui a obtenu une rallonge, Les signaux semblaient donc au vert. Mais la Hongrie et la Pologne, rejointes par la Slovénie, ont bloqué le processus, comme M. Mizzon l'a expliqué. Le point de blocage est connu : c'est leur opposition au mécanisme de conditionnalité au titre de l'État de droit. Ce point de blocage n'est pas une surprise. Comme le Sénat l'avait souligné dès sa première résolution sur le CFP, la mise en oeuvre d'une telle conditionnalité dans l'accès aux fonds européens suppose des critères objectifs et une méthode d'appréciation transparente. C'est aujourd'hui le coeur du sujet. Ce blocage devrait être évoqué aujourd'hui au Conseil européen. Hier, lors des questions d'actualité au Gouvernement, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes nous a indiqué que « des solutions pratiques pouvant passer par certaines clarifications techniques de ce mécanisme » étaient à l'étude. le secrétaire d'État, vous avez ajouté : « En dernier ressort, s'il le faut, nous regarderons comment avancer sans les pays qui bloquent, car l'Europe ne peut pas être retenue en otage par un certain nombre de gouvernements ne souhaitant pas respecter le socle essentiel de notre projet politique.

Monsieur le secrétaire d'État, je souhaite donc que vous nous éclairiez sur les solutions pratiques à l'étude et que vous nous confirmiez qu'en tout état de cause, il n'y aura pas de décalage dans la mise en oeuvre du CFP et du plan de relance français. Mais ce qui compte plus encore à mes yeux, c'est de partager de nouveau la conviction que le tout est plus grand que la somme des parties, que l'Europe, fondée sur des valeurs communes, porte un projet d'avenir que nous assumons collectivement un projet qui répond aux attentes et aux besoins de nos concitoyens en matière de sécurité, de gestion des frontières, de développement économique et social ; un projet qui répond aux défis actuels en matière de numérique et de lutte contre le changement climatique. Tel sera l'enjeu essentiel de la Conférence sur l'avenir de l'Europe.

que reviendra la responsabilité de ratifier la décision sur les ressources propres. C'est à nous que reviendra la responsabilité de permettre l'introduction de nouvelles ressources propres sur la feuille de route qui a été négociée.

Joly. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, avec une contribution annuelle de la France passant de 21,5 milliards d'euros à 26,9 milliards d'euros, nous sommes à un tournant dans l'effort financier de notre pays au budget de l'Union européenne.

; enfin, les conséquences de la crise économique liée à la pandémie, pour 1,6 milliard d'euros. En parallèle, nous nous trouvons à un tournant s'agissant du budget européen lui-même, avec le plan de relance européen, d'un montant de 750 milliards pour les trois années à venir, financé essentiellement par emprunt sur les marchés financiers. D'une part, au regard des problématiques du financement de ce plan, on ne peut que s'étonner que les négociations du Conseil européen n'aient pas sonné le glas des rabais sur la contribution au budget européen. permettent à certains pays de payer moins qu'ils ne devraient. Bien au contraire, pour satisfaire aux exigences des pays dits frugaux, qui- je le rappelle -ne représentent que 10 % de la population européenne, le Président de la République et la chancelière allemande ont accepté que ces rabais soient maintenus pour l'Allemagne et même fortement augmentés pour le Danemark, les Pays-Bas, l'Autriche et la Suède. Quel mauvais signal pour la solidarité en Europe, d'autant qu'il s'agit des pays les plus riches D'autre part, nous arrivons clairement aux limites d'un système : la question des ressources propres devient pressante pour permettre à l'Europe d'affronter les défis qui sont devant elle et assurer le remboursement de l'emprunt européen, principale source de financement du plan de relance. Il est désormais nécessaire de bâtir une véritable fiscalité européenne ! C'est aussi un enjeu de souveraineté. Pourquoi ne pas mettre en oeuvre immédiatement la taxation des géants du net qui ne paient pas d'impôt en Europe alors qu'ils réalisent la majeure partie de leurs profits sur le territoire européen ? une taxe sur les transactions financières, qui permettrait aussi de protéger notre système financier ? Ou une taxe carbone à nos frontières communes pour protéger nos productions Certes, les chefs d'État et de gouvernement s'y sont engagés lors du Conseil européen du 21 juillet dernier. Mais nous avons besoin de gages sur la rapidité de mise en oeuvre.

de programmes européens alors que le compromis entre les États membres avait été annoncé comme bouclé. Je me félicite spécialement des avancées obtenues par mes collègues sociaux-démocrates du Parlement européen, qui ont pesé de tout leur poids pour rééquilibrer ce compromis en faveur des priorités de nos concitoyens : la santé, le climat, la jeunesse et la culture. Pourtant, des inquiétudes et des interrogations demeurent. Les États membres ont procédé à des coupes massives dans tous les programmes européens stratégiques, dans le cadre du budget européen comme du plan de relance adossé. Les exemples ne manquent malheureusement pas, dans le domaine de l'industrie, avec la suppression de l'instrument de solvabilité destiné

destiné à attirer les investissements privés traditionnels sur garantie publique européenne en direction des infrastructures dites durables et de la numérisation, de la santé, des PME et du secteur social, a été finalement supprimée par les États membres le 4 novembre dernier. Comment ne pas évoquer aussi la ruralité, alors que les crédits pour le développement rural sont en forte régression ? C'est ne pas comprendre que la relance de l'Europe passe aussi par ces territoires, qui disposent d'un potentiel pour répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés en termes d'environnement, de santé et d'économie, De même, nous devons rester vigilants sur la progression de l'enveloppe consacrée à la politique agricole commune, qui, malgré le maintien de ses crédits, un moment menacés, ne satisfait complètement ni les agriculteurs, ni les organisations environnementales, ni les citoyens. ailleurs, nous devons continuer à lutter contre la sous-exécution chronique des crédits de cohésion. Elle représente près de deux années budgétaires de l'Union européenne ! La Cour des comptes européenne s'en est même inquiétée. Notre vigilance doit porter également sur l'articulation complexe des huit fonds de cohésion, dont les financements constituent potentiellement une contribution réelle à la relance de l'économie européenne, à la solidarité et à la cohésion

par la Pologne et la Hongrie, rejointes par la Slovénie, de la finalisation des accords sur le cadre financier pluriannuel et le plan de relance européens. Il est essentiel et urgent de désamorcer leur veto, lié à la conditionnalité de l'accès

la participation de la France au budget de l'Union européenne pour l'année 2021 est particulière à plusieurs égards. D'abord, nous faisons face depuis le mois de mars dernier à une crise sanitaire et économique d'une violence inouïe. Les pays européens adaptent sans cesse leurs mesures pour enrayer cette crise et protéger les citoyens européens des conséquences de la pandémie. L'Union européenne mobilise des moyens importants, notamment financiers et économiques. Je pense bien sûr à la première émission de dette commune par la Commission européenne au nom de l'Union européenne, à hauteur de 750 milliards d'euros. Celle-ci s'inscrit dans le budget de long terme de l'Union européenne. Ensuite, l'année 2021 sera le premier exercice du nouveau budget de long terme, le cadre financier pluriannuel 2021-2027. Les discussions sont en cours depuis 2018, et la crise sanitaire n'a pas simplifié les négociations. Lors de l'examen de la participation de la France au budget de l'Union européenne de l'an dernier, nous avions déjà alerté sur la complexité de trouver un accord équilibré, puissant et adapté aux objectifs nouveaux et historiques de l'Union je déplore que le CFP soit pris en otage par le veto de la Hongrie et de la Pologne, rejointes par la Slovénie. L'unanimité nécessaire est mise à l'épreuve du respect de l'État de droit comme condition du versement des fonds européens. C'est inadmissible je ne doute pas de l'énergie que vous déployez sur ce dossier. Je vous renouvelle notre confiance pour arriver le plus rapidement possible à une solution respectueuse de nos valeurs européennes. nous ne pouvons écarter ni l'éventualité que rien ne soit résolu avant la fin de l'année ni les menaces sur l'impossibilité d'adopter un budget européen pour 2021.

Quelle incidence prévoir sur le montant de cette dernière, qui a déjà augmenté de plusieurs milliards d'euros par rapport à 2020 ? La contribution des États membres n'étant pas la seule source budgétaire de l'Union européenne, quel effet aura la crise sur les autres recettes et sur l'exécution de la contribution française pour 2021, alors que la pandémie se poursuit ? Bien entendu, la crise à laquelle nous faisons face et les effets du Brexit nous demandent des efforts supplémentaires, auxquels nous sommes prêts. Mais nous sommes aussi conscients de l'exercice d'équilibriste que nous pratiquons. Pour illustrer mon propos, permettez-moi d'évoquer le plan de relance français, de 100 milliards d'euros, dont 40 % devraient être financés par l'instrument de relance européen, qui ne sera adopté qu'avec le cadre financier pluriannuel. Ces 40 milliards d'euros espérés ne seront évidemment pas automatiques, mais conditionnés au plan national de relance et de résilience que la France présentera à la Commission européenne, chargée de son évaluation.

collègues, si nous voulons répondre à la crise, effectuer notre transition écologique, engager notre évolution numérique, sécuriser nos frontières et notre territoire et prendre notre place dans les affaires du monde, nous avons besoin d'Europe et d'un budget solide.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, rappelons-nous un instant où nous en étions encore tout récemment : avec le Brexit, au plus fort de la crise sanitaire, on a pu penser que c'était fichu, que la désunion européenne était engagée.

donne : accroissement possible de la solidarité européenne ; affichage clair d'un large effort de relance ; et, je l'espère, concrétisation, impérieuse, de nos engagements climatiques. sur recettes que nous examinons pourrait passer pour la validation d'un simple chiffre, une information annuelle au Parlement sur l'estimation du montant dû par notre pays. L'article 31, c'est sobre, sec et précis : trois lignes pour 26,9 milliards d'euros. Pour nous, c'est un petit bout de soirée de débat. Or je crois que c'est bien plus que cela. Cette année, ce prélèvement est éloquent. Il concrétise l'accroissement de la solidarité européenne de l'Union européenne pour relancer ses économies et réaliser l'indispensable transition écologique. Ne débordons pas d'optimisme pour autant : on a avancé, mais ce n'est pas gagné. Les forces de fragmentation, les replis à courte vue font et feront encore des dégâts. Les mécanismes unanimitaires et les conditions de négociation interinstitutionnelle facilitent, on le sait, les blocages et les chantages. Les dirigeants actuels de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovénie risquent fort de nous ramener à la vieille recette des compromis paralysants. La frugalité dont se targuent certains est une façon élégante de désigner une pingrerie totalement inopportune face à l'importance des enjeux. Et que dire de ces fameux rabais des années 1980, qui survivent à leur disparition formelle, maintes fois annoncée ? Le prix à payer pour cet accord à vingt-sept n'est pas toujours bien reluisant, et l'intérêt budgétaire de la France a dû y laisser quelques plumes. Monsieur le secrétaire d'État, ne cédez pas plus, ne cédez pas trop ; ne perdons pas l'essentiel dans cette phase délicate. Un accord prometteur a été trouvé avec le Parlement européen : il s'agit de tenir pour que ces promesses se concrétisent. Tenir, c'est avancer résolument sur les ressources propres calendrier rapide à respecter et niveaux visés à maintenir. Le choix de l'endettement commun est celui d'un dessein partagé. C'est aussi l'obligation collective de dégager des ressources nouvelles et de modifier rapidement la donne budgétaire d'une Union ans après le traité de Rome, chacun pour soi fait encore le solde de ce qu'il verse et ce qu'il récupère, dans un calcul toujours faussé. Le chantier des ressources propres, c'est la seule et la bonne manière de casser ces logiques de copropriétaires crispés, « assis, genoux aux dents », comme dans le poème de Rimbaud Ces ressources propres seraient inopérantes si elles devaient être instaurées au rabais. Si la taxe plastique qui vient d'être mise en place est positive, elle n'est pas pour autant le modèle précurseur. D'ailleurs, il s'agit non pas d'une taxe, mais une nouvelle modalité de calcul des contributions nationales. Nous avons besoin de passer à tout autre chose : mécanisme carbone aux frontières, taxe sur les géants du numérique. Autant de leviers qui doivent faire bouger sérieusement les lignes des transitions nécessaires ! Il s'agit de faire en sorte que ceux qui tirent le plus de profits du marché européen contribuent à leur juste part à la chose publique et au bien commun. En clair, une taxe sur les transactions financières doit viser cinquante milliards d'euros à Les ressources propres peuvent être des moyens d'hâter la transition écologique et d'entraîner nos partenaires extérieurs dans ce mouvement. C'est la même logique qui doit de plus en plus présider à nos relations commerciales et aux accords commerciaux. Les accords de libre-échange sont désastreux s'ils ne s'inscrivent pas dans le respect des objectifs climatiques et de la trajectoire de l'accord de Paris ! Vous l'avez compris, le groupe écologiste votera cette contribution à l'effort européen. Vous pouvez compter sur son exigence pour que cette feuille de route, à la hauteur de la volonté du Parlement européen, tienne effectivement ses promesses

Nous connaissons tous la mécanique des rêves : un mélange de craintes, d'éléments réels et de fantasmes refoulés en journée, qu'agrège soudainement notre inconscient dans l'onirisme des ombres de la nuit. des ombres de la nuit. Dans mon cauchemar, la paisible galaxie Europe était soudainement percutée par un astre noir, une terrible pandémie portée par un virus inconnu déferlant sur tout notre continent, et bien au-delà. Une panique des populations attisée par de piètres prophètes de France et de Hollande, cet autre pays des faux mages, ... Quel poète ! ... conduisait notre pays à fermer ses frontières et à choisir de quitter l'Union européenne, le tout accompagné de surréelles scènes de « Frexiters » en liesse,

terrasserait le dragon. Cauchemar dans mon cauchemar : mon cerveau implosait en se demandant comment, à leur réveil, j'expliquerais à mes enfants qu'on venait d'assassiner leur avenir ; comment leur père, en quarante ans d'engagement européen, n'avait rien vu venir ; comment, en tant que parlementaire, il n'avait rien pu faire pour empêcher cela. Mon réveil en sursaut mit heureusement fin à cette ignominie. Après le choc, j'en revins donc aux affaires courantes et je m'attelai à la préparation de cette intervention. Que du bonheur, du moins, de la facilité, puisque voilà dix ans que je m'adonne tous les ans à cet exercice un brin répétitif ! Un simple copié-collé de mon discours de l'an passé aurait presque pu suffire. L'intitulé de l'article

Les raisons de cette augmentation de 5,9 milliards d'euros par rapport au montant exécuté en 2019 ont déjà été explicitées par les orateurs qui m'ont précédé. Je n'y reviens pas. que la somme est coquette et que ces nouvelles « poignées d'amour », certes séduisantes, touchent à notre portefeuille. Il est bon d'en avoir une pédagogie augmentée auprès de nos concitoyens, afin d'éviter les chimères malveillantes qui pourraient en résulter. Monsieur le secrétaire d'État, dans la période très difficile que nous et nos partenaires européens traversons, il est important de clamer haut et fort qu'on ne saurait rallumer les étoiles d'un drapeau européen un peu flétri avec de simples bouts de chandelles. Il est important de dire et de redire tous les bénéfices que notre pays tire de son appartenance à l'Union européenne, de manière directe ou indirecte, le plus souvent invisible, notamment au regard d'une comptabilité budgétaire qui ne rend pas compte des retours et externalités positives. Monsieur le secrétaire d'État, voilà des années que je réclame

en rendant imperceptibles ses qualités que nous en préserverons l'avenir ! La parole Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, crise sanitaire, Brexit, nouveau cadre financier pluriannuel : l'Union européenne est à la croisée des chemins, et dans des conditions difficiles. Reconnaissons qu'elle a choisi le cap de la solidarité. L'accord politique du mois de juillet dernier sur l'instrument de relance adossé au CFP est une étape majeure de l'intégration européenne, tout comme celle de l'amorce, la semaine dernière, d'une entente sur de nouvelles ressources propres. Le RDSE approuve pleinement cette évolution. Pour la France, avec un prélèvement européen en hausse de 25 % par rapport à 2020, l'article 31 traduit l'Europe que nous pouvons. En effet, l'effort financier de 26,9 milliards d'euros fait de la France l'un des premiers contributeurs nets. Compte tenu de ce niveau d'engagement, celui-ci doit aussi se traduire par l'Europe que nous voulons. Quelles doivent être nos priorités aujourd'hui ? Vous ne serez pas étonnés que notre groupe soit favorable à la recherche d'un équilibre entre politiques dites « traditionnelles » et nouvelles priorités. Nous nous réjouissons que la copie de 2018 de la Commission sur le budget de la PAC ait été revue à la hausse sur proposition du Conseil, avec 19,6 milliards d'euros supplémentaires. À l'époque, la diminution des moyens consacrés à l'agriculture était un sujet majeur d'inquiétude. L'Union européenne et, au sein de celle-ci, la France portent des ambitions pour notre agriculture qu'il faut concrétiser rapidement. Il ne s'agit pas seulement de protéger nos agriculteurs, soumis à une concurrence économique croissante. Il faut aussi s'atteler encore davantage à l'urgence climatique ; les exploitants y sont partie prenante. j'ai eu l'occasion de le rappeler ici, lors du débat à la suite du dernier Conseil européen, la proposition d'écorégime va dans le bon sens. Ce dispositif fait écho au Pacte vert pour l'Europe. Les agriculteurs qui s'engagent dans la transition écologique doivent être soutenus en priorité. priorité. Le volet environnemental ne doit pas occulter toutes les autres problématiques. Et elles sont nombreuses : revenus, compétitivité, filières, transmission ... Monsieur le secrétaire d'État, chaque État doit remettre un plan national stratégique de la PAC en début d'année prochaine. Où en sommes-nous ? J'en viens aux nouvelles priorités. Je saluerai en particulier l'ébauche d'une Europe de la santé, bien que la dotation de 3,4 milliards d'euros du CFP soit en retrait par rapport à 2018, y compris en tenant compte de la rallonge obtenue le 10 novembre dernier grâce à l'initiative du Parlement européen. Par ailleurs, les échéances me paraissent bien lointaines. La Commission veut muscler la gestion des crises sanitaires- mais seulement en 2023 ... -, avec la création de l'Autorité pour la réaction aux urgences sanitaires. Au regard de ce que nous venons de vivre avec la covid, serait de ne pas trop tarder, en particulier sur la mise en oeuvre d'une stratégie de souveraineté médicale. L'Europe ne produit plus de paracétamol. Est-ce bien raisonnable ? Enfin, les attentes sont nombreuses à l'égard de l'instrument de relance de 750 milliards d'euros. Je ne reviendrai pas sur le fond, si ce n'est pour regretter le rétrécissement de la part de subventions au profit des prêts. Certes, c'est le fruit d'un compromis avec les pays dits « frugaux ». Mais, pour la suite, gardons le cap de la solidarité, qui donne à l'Union européenne tout son sens. Le sens de l'Europe, c'est aussi le respect des valeurs démocratiques en son sein. À cet égard, quelle serait la réponse à l'attitude de blocage, pour ne pas dire de chantage, de la Pologne, de la Hongrie et, désormais, de la Slovénie si celle-ci devait persister ? Espérons que ces trois pays reviennent à la raison et qu'un voile ne soit pas jeté sur le respect de l'État de droit, condition forte à l'adhésion communautaire. En attendant, le RDSE, fidèle à son engagement européen, approuvera l'article 31 du projet de loi de finances. La parole

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la crise sanitaire en cours et le plan de relance consécutif, le Brexit et ses répercussions, bien tangibles sur le budget commun à venir, conjugués à la détermination en cours du cadre financier pluriannuel de l'Union pour les sept prochaines années

France. Le budget prévu au titre de la participation de la France au budget européen s'élève à 26,9 milliards d'euros, soit une hausse de 5,9 milliards d'euros par rapport à 2019 et de 3,5 milliards d'euros par rapport à la prévision revue de 2020. Cela représente environ 7,1 % des dépenses pour notre pays. ce budget, nous ne pouvons que donner notre blanc-seing, puisque la marge de manoeuvre de notre parlement est infiniment faible, voire inexistante, sans parler de l'enrobage très consensuel que le Gouvernement nous propose, alors que rien n'est encore entériné, les États membres peinant à s'harmoniser sur les conclusions de cet accord, de surcroît mis à l'arrêt par la Hongrie et la Pologne ce lundi pour des questions de respect de l'État de droit. Mais surtout, mes chers collègues, laissez-moi vous dire que ce plan de relance n'a rien d'historique.

Pourquoi pas, me direz-vous, puisque nous prônons l'Europe de la solidarité ? Certes, mais l'Europe de la solidarité ne doit pas être l'apanage de quelques États membres, quand d'autres, plutôt partisans d'une Europe des concurrences nationales, bénéficient de rabais exponentiels tout en continuant d'abriter de grands groupes adeptes du dumping social et et fiscal. Ainsi, l'Europe de l'argent persiste et signe. Pourtant, des solutions de financement pour avancer vers une union européenne en commun et solidaire existent. mentionnerai au moins deux importantes. La première consisterait à s'appuyer sur l'immense pouvoir de refinancement de la Banque centrale européenne, seul acteur à même de redonner aux États une marge de manoeuvre budgétaire plus que jamais nécessaire aujourd'hui.

Monsieur le secrétaire d'État, le Gouvernement s'honorerait à travailler à la tenue d'une conférence européenne sur la dette, afin d'en annuler une partie et de restructurer l'autre.

Cela est bien timide, trop timide, et plus que décevant eu égard à la création de la ressource propre qui permettrait à elle seule de financer le plan de relance-beaucoup de collègues l'ont évoquée-, à savoir la taxe sur les transactions financières.

Nous vivons une crise sanitaire économique sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Tout est à rebâtir, et les rouages du capitalisme financier sont trop bien huilés, trop bien gardés pour être empêchés par quelques grains de sable. Il faut s'en prendre au mécanisme même et à ceux qui l'activent. Ils sont nombreux et puissants. C'est pourquoi la réponse doit être considérable et intraitable.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la participation française au budget de l'Union européenne pour 2021 constitue à bien des égards un révélateur. un révélateur de crise, puisque sa forte augmentation est en grande partie un stigmate budgétaire du Brexit, mais aussi des conséquences de la crise sanitaire, au niveau tant des recettes que des dépenses. À situation exceptionnelle, moyens exceptionnels. un révélateur de cohésion puisque face à ces épreuves, les États membres avaient dans un premier temps fait le choix de maintenir le niveau global de leur ambition budgétaire commune, avant, dans un second temps, de mettre en oeuvre de manière conjointe un plan de relance économique à tout point de vue inédit.

l'habileté de certains États membres dans la négociation du cadre financier pluriannuel. Ainsi, les pays dits « frugaux » ont su tirer les marrons du feu budgétaire : ils ont non seulement conservé leurs rabais, mais sont parfois même parvenus à les augmenter. La France, d'une certaine façon affaiblie politiquement et économiquement, n'a pas été en mesure d'y faire obstacle. Elle paie peut-être aussi ses déficits du passé et l'image d'un pays qui n'a pas su ou pas voulu mener les réformes structurelles importantes. La France, dans sa grande générosité, sera le premier financeur en faveur de pays bénéficiant d'un revenu par habitant supérieur au nôtre ; c'est tout de même paradoxal Je regrette que la frugalité de ces pays ne contribuant pas autant à la sécurité collective et à la lutte contre le terrorisme les ait conduits notamment à réduire les crédits du Fonds européen de défense et les ambitions européennes spatiales.

y compris même après 2027. Ce revers budgétaire pour notre pays- car c'en est un -au regard des positions qu'il a défendues dans la négociation illustre par ailleurs une réalité objective qu'en tant que parlementaires, nous ne pouvons pas ignorer : l'envolée en l'envolée en 2021 de la contribution française n'est en rien conjoncturelle. Je ne méconnais rien des bénéfices économiques tout à fait considérables que nous procure notre appartenance au marché unique et à la zone euro, ainsi que notre participation aux politiques communes de l'Union. Mais les faits sont têtus : la France versera en moyenne 28 milliards d'euros par an durant les sept prochaines années, contre 20 milliards d'euros entre 2014 et 2020. C'est considérable

Cette préoccupation m'amène à m'interroger sur les modalités de financement du plan de relance préparé par les chefs d'État et de gouvernement. Nous ne sommes pas nécessairement opposés au principe de l'emprunt européen- cela s'est déjà pratiqué dans le passé, certes pour des volumes plus modestes -, mais mais la communication du Gouvernement sur le sujet se limite à annoncer que le plan européen financera notre plan de relance national à hauteur de 40 %.

intéressants, rien n'est vraiment expliqué sur la manière dont cet argent sera remboursé. Pour paraphraser- une fois n'est pas coutume -le Président de la République, il n'y a pas d'« argent magique ». Si la valse des milliards d'euros mobilisés ces derniers mois peut nous donner l'impression inverse, les sommes empruntées devront bien être remboursées, n'en déplaise à certains, certes pas directement par les États membres pour ce qui est du volet « subventions » de 390 milliards d'euros de la facilité pour la reprise et la résilience, mais par le budget de l'Union. Sans pouvoir préjuger des taux de croissance de chaque État membre dans les trente ans à venir, la part de la France dans le budget européen laisse entrevoir une participation au remboursement des emprunts

J'en viens à la question des ressources propres. L'accord politique global conclu entre le Conseil et le Parlement européen la semaine dernière contient une feuille de route détaillant l'introduction progressive d'ici à 2026 d'un panier de nouvelles ressources, dont certaines apparaissent de bon sens stratégique. Cet accord les prévoit, mais il ne les crée pas. Or les expériences de la taxe sur les transactions financières ou encore de l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés nous enseignent qu'en matière de fiscalité européenne, il y a généralement fort loin de la coupe aux lèvres. Rien ne garantit donc Rien ne garantit donc à 100 % que les engagements d'aujourd'hui déboucheront bien sur les ressources de demain. En tout état de cause, si ces nouvelles ressources propres devaient effectivement voir le jour, elles contribueraient à faire basculer le mode de financement de l'Union vers un tout autre modèle.

Si nous ne sommes pas, comme cela a pu être avancé un peu hâtivement après l'accord du 21 juillet, dans un « moment hamiltonien », force est de le constater, il s'agit tout de même d'un pas supplémentaire en direction d'un fédéralisme budgétaire qui ne dit pas son nom. Une telle évolution ne pourrait légitimement être gravée dans le marbre à la seule faveur de la riposte à la crise que nous devons affronter actuellement.

Enfin, il m'apparaît essentiel que les sommes mobilisées bénéficient à la croissance et à la compétitivité des pays de l'Union au travers de l'utilisation avisée des fonds octroyés, mais mais aussi du financement de réformes fondamentales qui devront assurer que l'argent emprunté par les Européens et gagé sur les finances des Européens bénéficie bien aux Européens et ne contribue pas seulement à alimenter l'économie de nos concurrents. Rien n'est moins sûr Je pense par exemple à la révision de nos règles de concurrence, au renforcement de notre exigence commerciale à tout niveau, au développement d'une politique industrielle et numérique offensive. Alors que les États-Unis, la Chine et d'autres pays

Elle doit aussi et avant tout se réformer et s'affirmer dans la cohésion face à des États puissances et à des entreprises mondialisées, qui, eux, ne font plus de politesse et avancent de concert.

nous examinons ce soir l'article 31 du projet de loi de finances pour 2021. Cette discussion intervient dans un contexte particulier à plusieurs titres. effet, 2021 constitue la première année du nouveau cadre financier pluriannuel européen, qui traduira les ambitions de la politique de l'Union européenne jusqu'en 2027. Mais l'année 2021 représente également un défi pour l'Europe, qui doit faire face à une crise sanitaire et, par voie de conséquence, à une crise économique sans précédent. Selon l'office statistique de l'Union européenne, la zone euro a enregistré entre avril et juin une baisse de 12,1 % de son PIB. Face aux nombreux enjeux, l'Union européenne a su répondre collectivement en réaffirmant son projet commun et en s'engageant à répondre d'une seule voix à la crise et aux immenses défis qu'elle doit relever. Le plan de relance et le choix de l'endettement communs sont des avancées inédites dans l'intégration et la solidarité européenne. Pour l'année 2021, la contribution française s'établira à 26,9 milliards d'euros, auxquels il faudra ajouter 1,6 milliard d'euros de droits de douane. Cela représente une hausse de 25 % par rapport à la loi de finances initiale de l'année 2020,

Cette augmentation tient à plusieurs facteurs : les conséquences de la crise sur les ressources propres traditionnelles de l'Union européenne, les augmentations des crédits de paiement, l'impact encore incertain du Brexit et les rabais négociés par certains États membres lors du Conseil de juillet dernier. Cette prévision reste soumise à des incertitudes. De plus, les négociations interinstitutionnelles ne sont pas terminées. Pourtant, nous ne pouvons que saluer l'accord trouvé le 10 novembre dernier avec le Parlement européen. Il entérine un complément budgétaire de 16 milliards d'euros appelé « ressources propres », sera réparti entre le programme Erasmus +, le programme de recherche Horizon Europe et le programme de santé, nécessaire pour poursuivre la lutte contre la pandémie actuelle. Cependant, la ratification de tous les parlements nationaux est nécessaire. Vous l'avez dit, la Hongrie, la Pologne et la Slovénie ont menacé de bloquer le processus si le versement des aides européennes restait conditionné au respect du principe de l'État de droit.

Malgré ces incertitudes, qui sont encore nombreuses, nous devons dire notre satisfaction s'agissant des nouvelles priorités de l'Union. Nous nous réjouissons du renforcement des objectifs le Conseil ayant porté de 25 % à 30 % les parts des dépenses totales du CFP et du plan de relance consacrées au climat. Cet effort budgétaire, en cohérence avec l'arsenal législatif annoncé par la Commission dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, dont la colonne vertébrale est la « loi climat

souligner la remise en oeuvre du chantier des ressources propres, nécessaires au remboursement de l'emprunt contracté pour le plan de relance. La première, c'est-à-dire la taxe sur les déchets plastiques non recyclés, doit être mise en oeuvre très prochainement. D'autres devraient suivre : la taxe sur les géants du numérique, une taxe carbone aux frontières et, à horizon plus lointain, une taxe sur les transactions financières. Si le calendrier établi par l'Europe semble précis, que se passera-t-il si nous faisons face à une absence de ressources suffisantes pour rembourser notre emprunt ? Les termes de l'accord de juillet dernier précisent bien que ce serait alors aux États membres de prendre le relais.

il ne faut pas occulter le fait qu'elle est également l'une des principales bénéficiaires des dépenses de l'Union. En 2019, les dépenses européennes au profit de la France se sont élevées à 15,1 milliards d'euros.

d'euros. Le plan de relance sera concentré sur le début de la programmation budgétaire. C'est donc un doublement du budget annuel de l'Union européenne qui est proposé

complète de notre plan de relance pour son montant intégral de 100 milliards d'euros. C'est essentiel pour nos entreprises, nos concitoyens et nos territoires. Pour autant, remboursement ne signifie pas soutien secondaire ou superflu : sans cette garantie de 40 milliards d'euros, nous n'aurions pas pu

Ces crédits arriveront, je l'espère, dès le premier semestre 2021. Il y a aujourd'hui un blocage, qui est lié à la question de l'État de droit. Comme je l'ai dit hier devant la Haute Assemblée, nous ne renoncerons pas à cette ambition de principe,

Il n'y a pas de finances publiques magiques, vous l'avez rappelé, mais il y a en revanche des iniquités ou des injustices fiscales à réparer. L'Europe progresse sur ce chemin. J'espère que nous pourrons en discuter dès l'an prochain pour franchir une nouvelle étape sur la mise en oeuvre de ces ressources.

l'avis du Gouvernement ?